La parole est à monsieur Patrice Joly pour une mise au point, au sujet d'un vote. Merci madame la présidente. Il s'agit du vote concernant le projet de loi relatif à l'accélération des processus des procédures liées aux nouvelles installations nucléaires. je voudrais que ce qui était considéré comme une non participation au vote. Soit aujourd'hui enfin maintenant. Prise en compte comme une abstention. Merci. La parole est à Madame, Jacqueline Eustache-Brinio également pour une mise au point, au sujet d'un vote. Merci madame la présidente, effectivement sur le scrutin public numéro 110, mes collègues Catherine Berluti Gilbert Favreau se Sylvie gouache avant Viviane Lopez Viviane Malet Alain Millon Albéric de Montgolfier Philippe pèse mec souhaiteraient voter pour mener la présidence. Si cher collègue. tu t'es donné de ces mises au point. Elles seront publiés au Journal officiel et figureront dans l'analyse politique. Les scrutins. La séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Dans la discussion des articles. Nous sommes parvenus à l'amendement numéro 72 rectifié au sein de l'Arctique. Le sept. Et nous sommes donc à l'amendement 72. Rectifié monsieur dessus. Merci madame la présidente. Cher collègue, Monsieur le Ministre, je suis content de vous retrouver parce qu'on a commencé à beaucoup. Débat sur l'article 7 et on avons ont besoin de vos éclairages parce que nous n'avons pas beaucoup avancé sur un certain nombre de garanties que nous demandions et nous l'avons dit, pour vous résumer les débats que cet article comporte un certain nombre de risques majeurs. Pour la vie privée et les libertés fondamentales. Nous ne souhaitons pas que ces mesures soient instaurées hein on va le répéter, c'est pourquoi nous avons proposé la suppression de cet article. Néanmoins il si elle venait quand même à être introduite Il est permis. Il est primordial de les accompagner de garanties pour mieux protéger. Nos libertés fondamentales et dans cet esprit de Concorde nous estimons indispensable. La transparence et l'accessibilité des algorithmes comme prérequis pour le contrôle démocratique de l'utilisation qui est faite de nos données de nos actes et liberté. Il nous apparaît comme légitime que le code source de l'algorithme soit accessible à toutes et tous celui travail dont celui-ci travaille hé apprends c'est la base de notre travail de contrôle. Il est également nécessaire d'empêcher la vente et la cession des données qui seront traités par ses algorithmes. Les pays occidentaux et la France ne fait pas exception malheureusement ont une longue tradition de commerce notamment en terme de matériel de sécurité avec des régimes beaucoup moins regardants sur les droits et des libertés et nous ne souhaitons pas que les données d'apprentissage de ces algorithmes collectés au moment des Jeux Olympiques mais aussi au moment de la Coupe du monde de rugby puissent être cédés ou vendus à des acteurs publics ou privés. Internationaux c'est une précision que nous jugeons fondamentales en termes de garantie universelle des libertés publiques libre accès des données est garantie éthique, voilà ce que nous proposons avec cet amendement. Si Monsieur dessus. Madame la rapporteure avis de la commission. Puisque c'est un débat, on a vu à propos de Parcoursup, on voit bien qu'en matière de sécurité, c'est quand même compliqué de rendre ouvert et accessible à tous des algorithmes qui sont destinées à nous protéger. Quant à inscrire la non-session des. Données d'apprentissage d'ores et déjà, c'est le cas, parce qu'elles seront effacées si elles n'ont pas eux donné de résultats et ensuite elles peuvent être conservées pendant un mois, mais uniquement pour s'entraîner. Ça reste sous la maîtrise de l'état, il n'y aura pas de session possible donc avis défavorable.

Évoquer 2 choses si nous rendons libre. Ces consultations d'algorithmes d'abord c'est une propriété industrielle. Et c'est un 1er point il faut quand même souligner qu'il est tout à fait normal qu'aucune entreprise de candidats. Si elle ne peut pas être propriétaire de son organisation technologique et deuxièmement surtout, argument qui devrait quand même vous frappez monsieur le sénateur, en tout cas l'hémicycle si nous rendons publics les algorithmes à des fins de sécurité. Les gens qui nous attaquent et terroristes et singulièrement les cyber terroriste. On a qu'à leur donner directement les clés du coffre et comment attaquer le camion, on ira beaucoup plus vite, puisqu'on va pas rendre publique la façon dont les algorithmes de sécurité. Serve évidemment à la protection pour une finalité particulière que sont les grands événements et singulièrement les Jeux olympiques. Sur le travail que font nos forces de sécurité à travers ses caméras. De vidéo protection, donc c'est évidemment un avis défavorable. Merci monsieur le ministre, une demande d'explication de vote monsieur dessus. Ensuite, vous venez de confirmer une partie de de de nos arguments que nous avons développées, que ces JO seront l'occasion pour un certain nombre d'industries de la sécurité d'emmagasiner à nombre de données d'enrichir. Leurs algorithmes pour pour plus tard, les revendent, y compris à l'international pour des régimes

l'Open source est une garantie de sécurité, y compris sur Internet. C'est par l'Open source et la collaboré la la collaboration des différents utilisateurs que nous avons renforcé, 100 de sécurité. Dans notre réseau internet je pense que, ouvrir ses algorithmes nous permettra à nous. En terme de parlementaires, d'avoir le, la compréhension suffisante pour voir qu'est-ce quelles quelles sont les informations qui sont collectées c'est important puisque nous avons un devoir de contrôle. Et puis, ça permettra aussi d'enrichir ses algorithmes pour les rendre effectivement plus efficace. Merci messieurs de ce Monsieur le Ministre. Je me suis dessus. Je propose qu'on on commence pas le débat en en faisant dire à l'interlocuteur, ce qu'il n'a pas dit donc je n'ai pas dit ce que vous avez dit, vous confondez 2 choses si je peux me permettre.

on ne garde aucune donnée elle revendue à personne parce qu'elles sont détruites et il a pas d'utilisation de données. Donc c'est pour cela que votre point est totalement satisfait ces données ne sont pas gardés ne sont pas vendus et deuxièmement il y a un processus industriels que sont les algorithmes et effectivement une entreprise. Oui, ce sera une entreprise, une entreprise a le droit de garder son processus industriel après vous dites c'est revendu et pour notamment des défunts qui ne sont pas démocratiques,

c'est exactement même chose que sur les caméras de vidéoprotection toute technologie, monsieur le sénateur, après la question, c'est ce qu'on veut être un État avec une technologie forte propriétaire de notre technologie à voir nos données à nous, la façon dont on a impose des industriels de fonctionner. Plutôt que de se faire imposer des cadres. Étrangers comme ceux des chinois se des Israéliens ceux des Américains et et d'autres pays encore, on préfère que ce soit une filière française. Oui avec des capitaux français que l'État peut regarder et peut considérer d'ailleurs que ils doivent être de d'intérêts vitaux que les services de renseignements peuvent regarder et ne ne pas être vendues. À la découpe, par exemple. Oui, il faut être fier des grandes entreprises françaises ça évite aujourd'hui si on avait eu la même raisonnement sont sur les moteurs de recherche, nous n'aurions pas sans doute Google aussi monopolistique et je vais appliquer vous êtes écologistes la même chose sur les panneaux solaires. Si on avait plutôt pris la révolution de des panneaux solaires, on n'aurait pas des panneaux solaires chinois, par exemple en France donc accompagner la législation mais tout le monde le sait, Monsieur le Sénateur accompagné la législation pour dire à nos industriels, voilà les finalités démocratique, dans un cas de d'état de droit, de sécurité comme les Jeux olympiques, ça nous évite de nous faire imposer des solutions dans quelques années différentes et effectivement ces solutions différentes, on le voit avec un certain nombre de scandales qui se sont nés et jamais avec des entreprises françaises. Vous l'aurez constaté, Pegasus. On est un bon exemple lorsque s'est développée avec un cadre français, hé bien nous pouvons parler aux industriels, on peut. Gérer en partie leurs actions les réguler regarder leur capital soyons fiers des entreprises françaises. Merci monsieur Ouzoulias. qui assure. L'analyse de de de l'algorithme et c'est ce qui se passe par exemple pour. Le contrôle des algorithmes des Gafam des des réseaux sociaux et la CNIL ne ne fait pas autrement. Donc ce que, ce qui serait intéressant, ça serait de, de mettre en place justement tout ce régime de contrôle des des algorithmes pour s'assurer. Ce qui a réellement dedans. Ce qui est ce qui est très regrettable. Monsieur le Ministre, c'est que s'agitant des des réseaux sociaux il y a une obligation de communication par la loi de ses algorithmes Elle n'est pas respectée, donc nos craintes sur les algorithmes de la vidéo sont. Rigoureusement les mêmes. Merci madame la présidente. Si cher collègue. S'il n'y a plus demandes d'explications de vote, je mets aux voix le 72 rectifié qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté et le 25 rectifié banalisation, c'est la banalisation de technologie et comme ce texte est un peu sensible que cet article 7 est un peu sensible, il nous paraissait utile que que le ministre de l'Intérieur puisse répondre à des questions qui garantissent qu'on s'engage dans un dispositif sécurisé. S'agissant des libertés publiques. L'amendement 23 rectifié vient apporter une précaution supplémentaire au stade du développement des logiciels d'Intelligence artificielle qui seront associés aux images vidéo. Le projet de loi prévoit que ces logiciels peuvent être développées directement par l'État ou par un prestataire extérieur qui choisit comme il s'agit de la première expérimentation du recours à l'Intelligence artificielle avec des enjeux dont on a dit depuis tout à l'heure qu'ils étaient extrêmement sensible. Nous pensons qu'il faut porter une attention particulière à la prévention des conflits d'intérêts. C'est pourquoi nous proposons de renforcer les exigences auxquelles le développement du traitement doit répondre si un fournisseur externe et choisi en prévoyant des garanties d'impartialité. En plus des garanties de compétences et de continuité d'activité qui sont déjà prévues par l'article 7, nous avons tenu compte des observations pertinentes comme toujours de la rapporteure pour que cette garantie d'impartialité se matérialise par une déclaration des intérêts détenus à date et au cours des 5 dernières années. Merci monsieur dur madame la rapporteure avis de la commission. Madame la présidente. Ce sera un avis favorable car nous pensons après des échanges que nous avons eu notamment en commission, que c'est une garantie supplémentaire qui va dans le sens du juste équilibre. Merci, monsieur le Ministre.

Oui nous allons voter cet amendement mais je voulais remercier ministre d'avoir en qui est en en quelques interventions. Conforter. Nos, nos, notre point de vue sur cet article qui n'est qu'un cavalier législatif destiné à faire en sorte que nos entreprises. Reprennent du départ de marché aux entreprises chinoises en terme de sécurité globale. Merci monsieur le ministre. Si cher collègue, Monsieur le Ministre. Mais Monsieur dessus pour le pour le bien-être de nos débats. Il peut pas y avoir de cavaliers législatifs, parce que c'est le texte initial du gouvernement, voilà je le dis pour le Conseil constitutionnel. Très bien, je vais mettre aux voix si vous le voulez bien le 23 rectifié qui a reçu 2 avis favorable. Qui est pour. Qui est contre.

D'autoriser l'utilisation de traitements algorithmiques en matière de vidéosurveillance soit prise après avis des assemblées délibérantes. Il nous semble s'agir d'une mesure de bon sens pour informer nos territoires des décisions qui sont prises des concernant le mécanisme de l'expérimentation est particulièrement intrusif et comporte des risques en matière de protection des données de droits fondamentaux aussi il ne paraît pas inapproprié d'associer les collectivités au processus décisionnel, d'autant que si l'utilisation du dispositif à vocation à rester relativement exceptionnel. Il ne semble pas que l'ajout de ce simple avis soit insurmontable du point de vue de la procédure. Merci. Merci cher collègue. Madame la rapporteure. Merci à la présidente. Ça sera un avis défavorable. Madame la vice-présidente. Nous sommes ici au Sénat, toujours très attaché à ce que les collectivités territoriales soient associés aux décisions et qu'il y ait un dialogue entre l'État et les collectivités. On l'a vu tout à l'heure sur l'organisation des manifestations et nous pensons que ce dialogue est nécessaire. Mais néanmoins, nous pensons que dans. La mise en oeuvre de de de procédures de sécurité. Telles que la vidéoprotection intelligente ce serait alourdir inutilement la procédure et que ça éviterait et ça rendrait difficile leur déclinaison opérationnelle sur les territoires d'autant plus que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales n'ont pas de compétences en matière de sécurité, c'est une compétence du maire. Avis défavorable. Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre. Oui puis je préciserai indépendamment des excellents arguments madame la rapporteure madame la sénatrice qu'il y a des groupements comme RATP SNCF qui ne font pas partie de l'assemblée délibérante donc rentrer votre amendement. Inacceptable Donc ce c'est évidemment un avis négatif.

Merci madame la présidente. Il nous paraît utile de rappeler que l'arrêté préfectoral autorisant l'emploi de du traitement algorithmique. À l'occasion d'une manifestation donnée précise le périmètre telle qu'il est strictement défini au paragraphe. 1 de l'article 7 à savoir le lieu accueillant la manifestation et ses abords, ainsi que les véhicules et en prise de transports publics et les voix desservant cet amendement vise à assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l'égard du public, ce qui est une condition indispensable pour permettre le déploiement de dispositif de caméras augmenter dans un climat de confiance à l'égard des autorités publiques. Si Monsieur Durand Madame la rapporteure avis de la commission. Merci madame la présidente. Ce sera un avis favorable. C'est un moment, précision utile. Monsieur le ministre. Hein je je mets aux voix le 24 qui a reçu 2 avis favorable qui est pour. Contre qui s'abstient. Il est adopté 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune le 62 monsieur dessus. Merci madame la la présidente. Il est précisé à l'alinéa 28 du présent article que dans certains cas, le public pourrait ne pas être informé de l'usage de caméras dites augmenter. Qu'est-ce qui pourrait bien légitimer une telle exception Monsieur le Ministre, qu'est qui justifierait que les citoyennes et les citoyens ne puisse pas avoir accès à des informations relatives à leurs droits et libertés. Visiblement nous ne sommes pas les seuls à trouver que les situations qui relèveraient de cette exception manque de clarté. La CNIL elles-mêmes s'interroge sur les les hypothèses dans lesquelles une telle exclusion s'avéreraient nécessaire elle recommande d'ailleurs que les conditions justifiant cette exclusion soit particulièrement limité. Or en l'état, aucune précision à ce sujet n'a été formulée par ce projet de loi. La CNIL estime dans son rapport sur le projet de loi que l'information des personnes de l'usage des caméras augmenter et je cite un élément essentiel pour assurer la loyauté des traitements dans un objectif de transparence à l'égard du public et qu'elle est indispensable pour permettre le déploiement des dispositifs dans un climat de confiance à l'égard des autorités publiques. Au groupe écologiste. Nous considérons que l'information du public est une garantie essentielle de la protection des droits et libertés des personnes et notamment du droit à la vie privée. Comment faire valoir ses droits d'opposition d'accès de rectification et d'effacement de ses données personnelles. Si on ne sait même pas que ces données existent à ce titre, nous proposons par cet amendement la suppression de cette dispense d'information du public de l'usage des caméras dites augmenter. Ah pardon excusez-moi chers collègues. Nous, on vous propose de compléter le travail utile de la commission qui a introduit une garantie supplémentaire pour assurer l'information du public sur l'emploi du traitement des données personnelles prévues par cet article 7, y compris lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entre en contradiction. Avec les objectifs poursuivis par le traitement donc dans ces cas, la Commission a prévu de renvoyer à une information générale organisée par le ministère de l'Intérieur. Je fais référence au paragraphe 2 bis nouveau inséré l'article 7 et si nous voulons que l'information du public soit pleinement appliquée, il convient de prévoir également dans la décision d'autorisation d'emploi prise par le préfet de département où le préfet de police à Paris que les motifs de dispense d'information du public soit accompagné a minima de l'information générale du public sur l'emploi du traitement algorithmique cette information nous semblait essentielle car elle conditionne le cas échéant la possibilité d'invoquer le respect du droit de personnes à l'égard de la bonne application de ces traitements de données personnelles. Augmenté par l'Intelligence artificielle sur le fondement du RGPD et de la directive. Police justice merci. merci. Si cher collègue. Avis de la commission. Merci à la présidente. Alors sur l'amendement 62 du sénateur dessus. Ce sera un avis défavorable. Pense que. Supprimer la possibilité d'exception au droit de l'information affaiblirait le dispositif et le rendrait beaucoup moins opérationnel. Et c'est la raison pour laquelle nous avions quand même. En commission des lois a ajouté une garantie sous la forme d'une information générale du public. Sur l'emploi des traitements algorithmiques. Organisée par le ministère de l'Intérieur pour informer les publics des enjeux concernant cette vidéoprotection. Intelligente. Donc ce sera un avis défavorable sur le 62 sur le 25 du Rhin qui renvoie cette information générale organisée par le ministère de l'Intérieur. C'est un avis favorable. Merci madame le rapporteur. Monsieur le ministre.

Les citoyens selon la volonté de de la CNIL et de la volonté du législateur qu'ils sont vidéo protégés ou vidéo surveiller le terme. Que vous souhaitez. On a eu ce débat pour sécurité globale sur d'autres sujets que les caméras de vidéoprotection. C'est effectivement comme vous l'avez très bien dit pour pouvoir être informé consulter les données personnelles qui nous concernent. Et puis évidemment si on le souhaite faire effacer. Ces données. Ce n'est pas pour être empêchés d'abord d'être filmés bien évidemment chacun le le comprendre. Mais l'Intelligence artificielle appliquée aux caméras de vidéoprotection avec. Qui qui est au au captation d'images ne vise pas à donner des éléments supplémentaires de séance des individus mais des situations que pourra faire très concrètement. Cette caméra dite Intelligence d'Intelligence elle pourra regarder quel est l'événement que nous souhaitons retrouver où la situation qui se sont retrouvés le comportement qui se sont retrouvés à rassemblement extrêmement intempestif.

de pouvoir retrouver des données qui lui sont personnelles mais l'Intelligence, ça c'est la caméra si j'ose dire classique qui le fait et qui le fait de manière générale et c'est pour ça qu'il me semblait que la vie était réservé pour votre un moment et finalement, si j'ose dire il ne mange pas de temps à votre, à un moment, c'est pour ça que je je le je le combat, pas plus que ça et sans doute est-ce l'avis positif qui a donné, madame la rapporteure. Mais l'information générale, elle est déjà donné par le ministère de l'Intérieur. Soit par les communes lorsqu'il s'agit de caméras ou là l'État l'État pour la préfecture de police évidemment de caméras déjà installées, chacun doit installer des panneaux publié dans le journal municipal. La présence de ces caméras y compris mobiles. Et tout autre type d'information, on a eu cette discussion pour les aéronefs et pour d'autres situations comme les drônes dans la loi sécurité globale mais en aucun cas. L'Intelligence artificielle ajoute quoique ce soit puisque. Il ne peut pas y avoir, il ne peut pas y avoir de captation. Sans caméra donc, cette information est déjà donné par la loi et l'Intelligence artificielle vise à retrouver des situations c'eût été extrêmement différents, si nous vous avions proposé la reconnaissance sociale. Qui la parle de sujet individuelle et donc évidemment l'information autour des données individuelles. Par ce moyen nouveau même dans un moyen de captation ancien aurait sans doute eu son sens de discussion. Donc vraiment je pense qu'il faut bien comprendre, pour ceux qui nous écoutent qu'il ne s'agit pas dans l'Intelligence artificielle de continuer à regarder des données personnelles, ce n'est pas ce que feront ces ces caméras. C'est des situations mais comme chacun a dû le voir sans doute dans des documentaires dans des films ou dans des reportages ou dans les auditions. Vous avez pu faire et ces situations sont extrêmement importantes. Imaginons que nous ayons à gérer une alerte à la bombe pour savoir si elle est sérieuse pas sérieuse qui a déposé le sac, dans quelles conditions il a déposé un sac. Est ce que cette. Situation ne dépose ça c'est un oubli ou c'est quelqu'un qui le fait de manière volontaire. Ça fait gagner énormément de temps au service de police qui l'a déposé en tant que telle, ou les personnes autour d'elle ne sont pas concernés par les les algorithmes et par la finalité que nous demandons législateur je constate d'ailleurs Monsieur dessus que est l'avis de la CNIL est l'avis du Conseil d'État. Sur un texte. Aussi complexes ont été sans réserve sur cette situation et les débats qu'on a eues précédemment et notamment sur la l'mise sur les questions d'image ou et tout c'était validé, vous l'aurez constaté par une excellente décision du Conseil constitutionnel dont je me réjouis donc je veux vraiment ici dire et je reçois le rapporteur Hervé qui a notamment évoqué ces sujets de données personnelles. Je voulais aussi dire encore une fois que la Haute Assemblée droit et rejeté l'amendement de Monsieur dessus pour confusion s'il ne faut pas me le permettez. Et voilà, la maman de ce dur hein. Sans doute est superfétatoire mais je veux bien donner un avis neutre. C'est-à-dire réservées pour l'adoption. C'est une sagesse Monsieur le ministre un avis défavorable. Sagesse neutre. Bon bah écoutez nous innovons aujourd'hui mais bon. Alors je mets aux voix. Ah pardon monsieur de support. Explications de vote et madame arriver. Merci madame la présidente, là on constate qu'on est en train de reculer sur sur un certain nombre de droits. Liés au à nos données à nos comportements. Vous venez de le dire, ces caméras enfin ses caméras elles existent, elles sont déjà là on va aller, on va leur ajouter un système qui va permettre de faire la différence entre différents comportements différentes situations. Qu'est-ce qui nous fait basculer dans une société de surveillance, c'est qu'un hein comporte un individu vous moi un autre. Va se trouver dans une situation sans ça, sans savoir ce que la caméra va chercher à contrôler dans ce comportement. Vous l'avez cité un oubli de sacs. Alors vous vous êtes rattrapés en disant que ce sera pas une donnée personnelle mais que ça peut faciliter quand même d'identifier la personne qui l'a oublié. Donc on est déjà en train de reculer un peu là-dessus. Bien sûr que si on est en train déjà reculé sur les les les comportements accepter question la Corse non acceptées qui définit a effectivement là on ne le sait pas ça sera défini dans les algorithmes, que vous n'avez pas voulu ouvrir. Donc on est en train de reculer sur un certain nombre de de droits et libertés et de la façon dont on peut nous individus protester conte la collecte d'un centre de données ensuite monsieur ministe je vous trouve extrêmement rigoureux sur le, la question des droits et libertés. Vous l'aviez été le 22 octobre devant devant nous que vous aviez présenté le dispositif de sécurité. Vous aviez dit le ministère de l'Intérieur n'utilisera pas de dispositifs. Illégaux qui n'ont pas été légalisée mais par contre un certain nombre de collectivités les utilisent déjà ces sont vos mots. Elle a su, vous n'aviez. Pas répondu ensuite à savoir quelles sont les collectivités qui utilise tout ça dans des quelques quelle est l'action du ministère de l'Intérieur pour lutter contre 8 usage abusif de ces technologies. On a déjà pu voir un certain nombre de marchés publics passés pour des technologies qui ne sont pas encore légaliser et donc j'aimerais bien leur réponse aussi là- dessus, vous qui êtes si respectueux du droit. Si cher collègue Madame. Simplement pour dire que cet amendement que que nous proposons et qui a été qui a un avis favorable de la rapporteure. C'est c'est pas quelque chose qui qui n'est anodin non plus. C'est-à-dire que c'est il s'agit pas d'une, d'une information individualisée, mais il s'agit de lier la décision à l'information c'est tout et donc je pense que ça permet plus de transparence, ça permet d'être plus clair. Alors vous avez dit ça mange pas de pain. Je crois que non en tout cas mais en tout cas, en tout cas ça ça fixe ça fixe les choses et ça officialise cette dimension de de l'information du public. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Je ne veux pas laisser monsieur dessus mais très rapidement faire croire que Moussa intérieur connaîtraient des situations illégales interviendrait pas. Non mais je suis respectueux. Là je suis surtout respectueux de la Constitution monsieur sénateur et en tant que représentants des collectivités locales, vous seriez très sourcilleux que l'article 72 de la Constitution soit respectée par le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que ces gens ont une compétence propre. Ne vous en déplaise des communes que de gérer la sécurité de leurs concitoyens en ce qui concerne la salubrité publique la tranquillité publique et les caméras de vidéoprotection et je pense qu'il y a un certain nombre d'élus écologistes qui serait bien inspiré d'appliquer les règles de la République le législateur leur a accordé, mais c'est un autre débat, c'est un autre débat, on en connaît quelques quelques collègues quelques collectivités locales qui en font eux-, mêmes revendications d'ailleurs on voit que c'est souvent là où la délinquance et parfois la plus importante, on aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez, appartient justement il appartient justement au tiers de confiance, évoquée par votre collègue. Communiste que de faire ces contrôles et je sais que la CNIL. Il est particulièrement attentif, donc ce n'est pas au ministère de l'Intérieur que de fait apporter une tutelle ça n'existe plus depuis 1981. Ça n'existe plus de 1980. Donc il faut être respectueux de la Constitution et l'héritage mitterrandien. Alors. Monsieur dur hein. Vous avez la parole. Une une explication de vote non pas pour allonger les débats mais pour préciser un point de vue politique. Très très cher à notre groupe au coeur de ce débat. L'argument de notre collègue dessus s'entend parfaitement. On comprend les réserves que son groupe peut avoir d'où d'ailleurs des des motions. Préalables. Nous considérer des ronds pour ce qui nous concerne. Qu'il existe un risque. De développement rampant à bas bruit d'un certain nombre de technologies. Et quand nous proposons qu'on puisse. En tant que législateur, s'intéresser à ces sujets fixer un cadre c'est pas pour autoriser ces technologies. C'est précisément pour dire dans quelles conditions. Alors même qu'elle s'invite partout dans nos vies personnelles et collectives. À quelles conditions peut les utiliser et pour avoir travaillé, ça a été rappelé plusieurs fois dans la journée avec Arnaud de Belenet et Marc-Philippe Daubresse sur la reconnaissance faciale. On voit bien qu'en plus qu'il y a une porosité des usages. C'est-à-dire que les citoyens consommateurs. Autorise dans leur comportement individuel, comportant en personnel, des choses qu'il réfute en tant que citoyen vis-à-vis de l'État et du coup il faut quand même résoudre ces tensions. Donc quand on propose. De légiférer de poser un cadre de définir des lignes rouges de temps en temps d'autoriser des expérimentations et c'est la démarche que notre groupe a, en l'espèce ça de son, de la surveillance intelligente c'est pas par plaisir de permettre tout et n'importe quoi. C'est au contraire pour que le carbone dans lequel c'était sont développés soit respectueux des libertés. Ah donc c'est vraiment l'esprit qui nous anime et d'où les les les amendements que nous avons déposée pour que l'information soit clair que les périmètres soit fixé que les durées soient limitées que les durées de conservation soient elles-mêmes limitées et qu'on puisse avancer ensemble dans la confiance vers l'usage de sa technologie. Merci cher collègue. Il n'y a plus de demandes de parole. Je vais donc mettre aux voix, tout d'abord l'amendement 62 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté et le 25 rectifié qui a reçu un avis favorable de la commission et une sagesse. Neutre. Du gouvernement. Qui est. Qui Qui est contre. Qui s'abstient les adopter. Nous passons à l'amendement 26 Monsieur dur hein. Alors on va connecter beaucoup de données, des données qui sont utiles, d'autres qui ne le sont pas. Ce que nous souhaitons au travers de cet amendement, c'est de préciser expressément que les données qui ne sont, qui sont considérés comme non pertinentes non adéquate et non représentative puisse être immédiatement supprimé sans attendent l'expiration du délai autorisé en commission, madame la rapporteure nous a fait observer que cette mesure est satisfaite mais il nous semble qu'elle apparaît pas clairement dans le dispositif de l'article 7 qui, au moment où nous parlons, est encore au stade de l'expérimentation. S'agissant d'opter pour la première fois, un dispositif inédit. On l'a vu qu'il est porteur d'enjeux nouveaux pour les droits, liberté qui est sensible. Le Sénat doit veiller à ce que figure dans la loi, les principes essentiels qui détermine l'usage des caméras augmenter c'est d'une condition qui pour nous est essentiel. Elle nous il nous semble qu'elle doit être explicitement mentionné. Le président de la CNIL d'ailleurs vient de s'exprimer sur le sujet et a rappelé que le principe de base de cette application et de conserver le moins longtemps possible les données. Si la CNIL veillera à ce que les données soient supprimées lorsqu'elles doivent-elles être autant inscrire dans le corps de la loi. madame la rapporteure avis de la commission. Oui merci à la présidente ce sera un avis défavorable. Il a été il était satisfait puisque ces données sont immédiatement détruite. Dès lors que elle. Elle devrait pas exister, pardon, donc on ne voit pas l'intérêt de le rajouter dans le texte. Je mais aux voix l'amendement 26 qui a reçu 2 avis défavorables qui est. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 27. Monsieur renonce à raser. Nina Simone à la présidente. Nous souhaitons lever une ambiguïté qui existe dans le texte entre 2 notions qui peuvent converger mais qui ne se confondent pas. La pluridisciplinarité et l'indépendance. C'est une bonne chose de prévoir que plusieurs spécialistes s'associent pour procéder à l'évaluation des caméras augmenter chacun travaillant dans son Champ d'application où sa discipline avec la méthodologie qui lui est propre. Nous sommes tout à fait favorable à cette optimisation des approches pour tirer les meilleures conclusions de l'expérimentation prévoir la meilleure communication possible entre les savoirs ne garantit pas l'indépendance du rapport final. C'est la raison pour laquelle, conformément à la recommandation de la CNIL nous souhaitons préciser que l'évaluation de l'expérimentation soit conduite en association avec des experts indépendants. Ce sera madame la présidente. Un avis défavorable. Nous pensons effectivement que c'est déjà prévu que ce soit. Des personnalités au caractère pluridisciplinaire qui a qui fasse l'évaluation pardon de l'expérimentation. Nous avons vu que et déjà eu des échanges sur le fait que cette expérimentation elle allait conduire sur une véritable évaluation qui permettra d'éclairer le législateur pour savoir s'il faut pérenniser ou non systèmes de vidéoprotection et que nombre de garanties ont été mises. Est introduite. Que ce soit un texte original ou que ce soit par la commission des lois pour que cette évaluation soit faite de manière la plus indépendante possible. Merci Monsieur le Ministre.

J'ai été saisi d'une demande de scrutin. Ah pardon monsieur dessus. nous ne. Considérons pas que les nos libertés publiques soit sujet à expérimentation y compris bornée dans le temps, nous considérons que cet article n'a rien à faire dans ce projet de loi n'en déplaise à Monsieur le Ministre, nous pensons qu'il est lié plus forme d'opportunisme sécuritaire destinée à marquer à masquer un certain nombre de défaillances, que le ministre a connu lors de de de de du fiasco du Stade de France. Et et donc nous, nous allons nous opposer à à cet article aucune garantie que nous avons proposé n'ont été acceptés et donc nous allons basculer via cet article, dans une, un nouveau régime de surveillance. Donc nous allons voter contre. Plus de demandes d'. Le j'été saisi d'une demande de scrutin public par les groupe écologiste solidarité et territoires et groupes républicains sur l'article 7 il va être procédé au scrutin public dans les conditions.

Sun ne demande à voter. Le scrutin est clos. Zulte sur ce scrutin. Nombre de votants 343 exprimés, 270. Pour, 243 contre. L'article est adopté. Un article additionnel après l'article sept. Un amendement numéro 3 présenté par Madame Eustache-Brinio, Merci madame la présidente. Je voudrais aborder les pneumatiques. D'aéroports de Roissy qui se trouve dans mon département pour préciser que face à la difficulté de lutter efficacement contre la multiplication des infractions de prise en charge illégale des clients par des trains public particulier des VTC ou des taxis clandestins. L'usage des images issues des systèmes de vidéoprotection, permettrait de renforcer la sécurité des voyageurs et la capacité des autorités judiciaires à déceler et qualifier ces infractions identifier les auteurs et accroître l'efficacité des poursuites lorsque celles-ci sont engagés. Cet amendement de bon sens signée par une soixantaine de sénateurs visant à permettre aux services compétents de l'État d'accéder plus simplement aux images facilitant l'engagement de poursuites vis-à-vis des contrevenants, participant ainsi à renforcer la sécurité des voyageurs à leur arrivée en dissuadant la pratique du racolage Qui vont celles et ceux qui vont à Roissy peut le constater. Quotidiennement. Les aéroports internationaux sont effectivement les principales portes d'entrée des voyageurs étrangers garde en mémoire que ce phénomène qui est une spécificité française, il faut le dire, porte atteinte à l'image de la France auprès des voyageurs et plus grand maman à la qualité d'accueil dans la destination tout spécifiquement lors des grands événements internationaux à venir et en particulier pour les JO et la Coupe du monde de rugby. Merci cher collègue. Madame la rapporteure avis de la commission. de pouvoir régler cette difficulté de VTC qui racolent. Dans les aéroports et notamment à Roissy, nous avons eu l'occasion souvent d'échanger sur ce sujet, mais malheureusement, chers collègues. Effectivement, c'est un vrai problème mais malheureusement chers collègues ce dispositif tel que vous le proposez n'est pas opérationnel. En effet, ce n'est pas le relevé de la plaque d'immatriculation du véhicule VTC qui suffira à constater l'infraction. Il faut être sûr qu'il n'y a pas eu de réservation préalable et donc c'est assez complexe à mettre en place via le système de vidéoprotection. En plus, c'est ouvrir une nouvelle finalité sur la vidéoprotection. Ça, pas sûr que ce texte soit le bon véhicule, même si nous comprenons chers collègues véritablement les enjeux et votre engagement sur ce sujet.

je voudrais quand même préciser que. Ces personnes qui viennent prendre les bagages. Des voyageurs qui arrivent, qui viennent les harceler qu'ils emmènent presque de force dans la voiture, par définition, ils ne sont pas réservés par définition parce que les VTC qui sont réservés, ils envoient des SMS à leurs clients qui les attendent un endroit précis et dehors donc voilà il faut juste relativiser les propos d'Alain là reporteurs que je respecte mais enfin ces gens qui viennent harceler les les les voyageurs à l'arrivée à Roissy et bien évidemment ce sont des gens qui viennent

madame de La Gontrie, vous avez la parole. Merci madame la présidente, simplement je je suis un peu comment dire perplexe et et interrogative face à cet amendement parce que. J'avais déposé avec mon groupe des amendements concernant l'organisation des transports publics. En Île-de-France et il a été. Opposé l'Arctique 45 célèbres dans cette maison notamment et donc ces amendements n'ont pas pu venir en discussion c'était concernant le la date d'ouverture. À la concurrence des réseaux de transport en commun de bus en Île-de-France qui ne promettent de joyeux mouvement de désordre éventuel si le gouvernement ne se décide pas reporter sa date de mise en en vigueur et. 45 dans ce cas-là. On se plie devant cette disposition et je vois que l'amendement de Madame Eustache-Brinio a été. Accepté donc peut-être que Madame la rapporteure, vous pourriez m'éclairer. Pourquoi les transports sont acceptées pour les uns. Et pas pour les autres. Madame la rapporteure. Vous avez la parole. La présidente. Madame la sénatrice de La Gontrie. Ici c'est bien différent parce que certes il y a une le sujet concerne les transports, mais ça concerne surtout la vidéoprotection. Or la vidéoprotection, hé bien dans le texte. Et là, l'amendement de Madame Eustache-Brinio visait bien l'article L 252 2 du code de sécurité intérieur donc il y a un lien Direct, ce qui n'était pas le cas, je suis désolé de votre amendement.

Oui madame la présidente. Merci, monsieur le Ministre, madame la rapporteure chers collègues un amendement qui vise à renforcer les mesures relatives aux enquêtes administratives de sécurité dans les transports. Compte tenu des enjeux sécuritaires liées aux JO. Les opérateurs de transport. Sollicite des enquêtes administratives avant tout recrutement ou toute mobilité sur un poste sensible au sein de leur structure. Néanmoins, afin de garantir une plus grande sécurité les nécessaire d'aménager les conséquences d'un avis d'incompatibilité rendue par le Service national des enquêtes administratives de sécurité dans le cas d'une mobilité d'un poste sensible. Vers un autre poste. Pendant la période des Jeux olympiques. actuel en l'état actuel, même en cas d'avis d'incompatibilité du SN EAS dans le cas d'une mobilité vers un poste sensible d'un agent RATP par exemple déjà affecté à une fonction sensible la personne concernée doit être maintenu sur son poste d'origine. Ce maintien constitue un risque important compte tenu de sa potentielle dangerosité reconnue, il apparaît totalement inopportun de reclasser sur le même périmètre sensible une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens et je pense notamment aux personnes fichées S. Merci cher collègue. Madame la rapporteure. Vous avez la parole. Oui merci madame la présidente ce sera. Cher collègue, une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable car nous pensons que votre amendement est déjà satisfait. En effet, l'article L 114 2 du code de la sécurité intérieure prévoit déjà que. La personne l'agent ne bénéficient pas. De l'autorisation préalable lié au criblage, hé bien il suite à l'enquête administrative pour être complète. Il peut être reclassés sur un poste et s'si le refus ce reclassement il pourra faire l'objet d'une procédure de licenciement qui n'a pas d'obligation de le maintenir sur ce poste censé puisqu'il n'a pas les autorisations, mais il y a une obligation de reclassement qui est déjà prévu et à défaut un licenciement. Merci madame la rapporteure. Monsieur le Ministre. Je vous remercie monsieur Tabarot. Vous avez la parole. Oui madame la présidente, je vais retirer cet amendement même si je peux entendre. Vos arguments au regard du droit du travail, notamment les opérateurs de transport ne sont pas des entreprises comme les autres, elles sont exposés au public très exposés aux risques les postes sensibles sont sur toutes les strates de l'organigramme, assurer la sécurité c'est aussi leur permettent d'assurer une meilleure protection de leur structure et faciliter le reclassement sur des postes non-sensible pour des emplois clairement identifié comme dangereux, car l'état actuel doivent être placés sur un périmètre qui reste quand même sensible. Mais je vais retirer car je vous apprécie beaucoup Madame la rapporteure se. Voilà cet amendement. Merci cher collègue. Et l'amendement 90 rectifié et retiré. Nous passons à l'amendement 91 rectifié monsieur Tabarot. Celui-là je vous préviens je vous apprécie beaucoup mais je ne vais pas le retirer. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, Madame la la rapporteure, chers collègues. Un autre amendement pour renforcer les mesures relatives aux enquêtes administratives de sécurité dans les transports en l'état actuel, seuls les salariés des entreprises de transport ou des gestionnaires d'infrastructures peuvent faire l'objet d'une enquête, même s'ils sont affectés à des postes sensibles au sein de la RATP par exemple les intérimaires sont juridiquement salariée de l'agence d'intérim. La RATP ne peut donc. Sollicité d'enquête administrative, c'est la même chose pour la SNCF qu'aurait corrélativement l'agence d'intérim n'a pas la possibilité de solliciter une enquête auprès du S. N. EAS puisqu'elle n'est ni une entreprise de transports publics de personne, ni une entreprise gestionnaire d'infrastructure, cet amendement vise donc à permettre aux agences d'intérim pendant la période des JO avant. Toute affectation sur des postes sensibles de solliciter elles-mêmes cette enquête. Si cher collègue Madame la rapporteure. un trou dans la raquette, entre guillemets si vous pouvez me passer l'expression, mais effectivement on voit bien que aujourd'hui les entreprises. De transport ne peuvent pas criblés les intérimaires Pas autorisé par la loi, donc il convenait de trouver un dispositif. Vous l'avez introduit pour au moins la période des JO via votre amendement et je pense que ça comble un besoin et donc c'est pour ça que je rendrai un avis favorable. Si Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre. je vous remercie monsieur Tabarot. Je voudrais bien sûr remercier Madame la rapporteure sur cet avis favorable, Monsieur le Ministre également et vous dire sincèrement que je pense qu'il faudra pérenniser cette mesure après les Jeux olympiques, Monsieur le Ministre, je vous le dis très clairement, je pense que ce sera indispensable pour autant, je garde l'amendement telle qu'il a été rédigé pour la période spécifique des Jeux olympiques. Merci. Merci, chers collègues, je vais donc mettre aux voix l'amendement 91 rectifié qui a reçu 2 avis favorable qui est pour. Qui est contre. Ça Pierre il est adopté. Nous en venons. Aux articles 9 10 et 11 appeler en priorité. Je mets aux voix l'article 9 qui. Pour. qui est contre. C'est le sien, il est adopté. Article 10, amendement 49 présenté. Monsieur Bakhit pardon. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre par notre amendement nous souhaitons supprimer l'article 10 du projet de loi qui prévoit l'élargissement de la procédure de criblage au fan zones et aux participants aux spectateurs des grands événements. Ce dispositif devrait conduire les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques prendre après autant d'enquêtes administratives. Près de 750.000 décisions relatives à l'accès des personnes et autres spectateurs aux installations équipements dans lesquels se dérouleront où seront retransmis les événements nous considérons qu'il s'agit manifestement d'une atteinte au droit fondamental d'aller et venir, ainsi qu'au droit à la vie privée et ce bien que l'administration émettent un avis conforme. Je vous remercie. Merci cher collègue. Avis de la commission, madame la rapporteure.

Étendue aux fans zones et aux participants. Or spectateurs de grands événements. Nous pensons que. Ces dispositions sont nécessaires pour assurer la sécurisation donc nous serons opposés. C'est un avis défavorable. Je vous remercie Monsieur le Ministre.

Est importante pour la sécurité de nos concitoyens. Puisqu'il faut bien imaginer que la cérémonie. Des Jeux olympiques, si je ne prends que celle-ci. C'est. 600.000 personnes peut-être plus. À Paris, sur 6 kilomètres le long de la Seine. Des kilos de Chebba Trocadéro les ponts. Et c'est aussi très certainement à Paris. Mais même en dehors de Paris dans toute la France. Des premiers jour des fans zones. Des écrans géants seront installés sans doute dans beaucoup de communes et c'est heures et on va voir des milliers de personnes des centaines et milliers peut-être plus d'avantage à Paris je vois qui voudront suivre la cérémonie d'ouverture et puis ensuite les grands événements de des Jeux olympiques. Et il y aura peut être additionnel m'en plus de monde dans l'ensemble de ses fans zones que. Dans le stade même dans la piscine même évidemment peut-être même. Que sur la CMU Arthur physiquement. Et si nous retirons la possibilité pour les services du ministère de l'Intérieur de criblé autant que nous le faisons dans des. Stades dont on a vu, nous avons vu, Monsieur le Sénateur. Dans le passé qu'ils étaient des lieux évidemment choisi pour être des attaques terroristes, alors nous laissons une un énorme Champ d'action possibles pour les terroristes de s'infiltrer et de commettre des actes. Contraires évidemment à ce que vous souhaitez, à ce que nous souhaitons et donc il s'agit pas de faire du criblage pour des criblage c'est-à-dire pour cela que ce texte s'inspire directement de ce que vous nous avez déjà autorisé sur les grands événements, d'ailleurs je vous rappelle que un grand événement et qualifiée comme telle par le ministre de l'Intérieur. Je prends un décret spécifique à ce qu'il a voulu le législateur et de je ne justifie pour justement prendre ces mesures. De criblage et évidemment personne ne peut nier que ce qui fera par 1 milliard 2 milliards, 3 milliards de personnes. Les Jeux olympiques, ce qui fera venir des dizaines de milliers de personnes dans des zones ne mérite pas ce tribunal, je suis vraiment c'est, c'est pas un argument d'autorité. Je crois que le groupe communiste devrait retirer cet amendement sinon un avis défavorable. Merci monsieur le ministre, s'il n'y a pas d'explication de vote je mets aux voix l'amendement 49 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour.

Merci madame la présidente. L'article 10. Donc on l'a vue modifient de façon pérenne les conditions d'accès aux grands événements en conditionnant les accès pour les sportifs, les équipes médicales, les équipes travaillant dans ces événements à la réalisation d'une enquête administrative. Si on peut considérer, on a entendu le Ministre une certaine justification sur des événements d'ampleur telle que les Jeux olympiques et paralympiques qui peuvent comporter des risques comme la cérémonie d'ouverture. Et qui peuvent justifier des modalités exceptionnelles pour la sécurité des personnes et des biens. Le présent article a vocation à s'appliquer en dehors des Jeux olympiques et paralympiques et à l'ensemble des grands événements et grands rassemblements de personnes. Le périmètre retenu pour les lieux susceptibles d'être visés par cette nouvelle procédure et large en sortent des espaces destinés à l'usage de tous voix publique lieux ouverts au public Parcs transports collectifs commerce le nombre de personnes visées par cette enquête administrative et large les acteurs, les sportifs, leurs équipes, les entraîneurs, les médecins, les kinés, les arbitres les chronométreurs en fait toute personne à l'exception des spectateurs serait soumise à une enquête administrative préalable selon la CNIL dans son avis du 22 décembre 2022. Une telle évolution conduirait à visée environ 50 à 60.000 participants pour les seuls jeux olympiques et paralympiques. Or, le gouvernement n'a transmis aucun élément justifiant un tel élargissement des périmètres et n'a pas motivé la pérennisation de cette mesure en fait à la réalisation de ces enquêtes administratives applique un traitement des données à caractère personnel ainsi que la consultation de certains fichiers dits de police ces données peuvent être conservées pour une durée de 5 ans au sein du fichier automatisation de la consultation centralisée des renseignements et des données sur ce point aucune garantie. Il a été mis en place pour que l'automatisation des consultations des fichiers concernés 2 conduisent pas à ce que des avis ou des décisions résulte de la seule inscription d'une personne dans un traitement de données à caractère personnel. La CNIL a alerté sur des possibles le préjudice important pour les personnes concernées par avis ou décisions défavorables défavorables à la suite de ses consultations pour l'ensemble de ces raisons nous demandant à ce que la mesure qui les dit proportionnée dit de garantit le respect des libertés individuelles soit supprimé et que ces deux alinéas soit donc supprimé de l'article 10. Ah pardon excusez-moi, discussion commune si je fais une erreur, Monsieur. Monsieur entraîne sur le 28. Oui merci madame la présidente, en fait une une nouvelle fois, nous tenons à dénoncer la stratégie cheval de Troie adoptée par le projet de loi qui prend prétexte de l'organisation exceptionnelle des Jeux olympiques et paralympiques pour envisager de modifier des dispositions problématique de manière pérenne. L'article 10 du projet de loi en off l'illustration. En ajoutant les participants aux personnes dont l'accès est subordonnée à une autorisation de l'organisateur délivré après enquête préalable de l'autorité administrative, soit l'intégralité des personnes accédant lieu concernant quel que soit leur statut et leur fonction en l'espèce une telle évolution conduira à élargir de manière très substantielle le périmètre des personnes concernées par ces dispositions, l'étude d'impact évalue cette extension du dispositif à 50.000 voire 60.000 participants pour les seuls jeux olympiques et paralympiques 2024 nous pouvons concevoir que cet élargissement du périmètre de l'enquête administrative est justifiée pour assurer la sécurité publique pendant la période des des Jeux olympiques dans un contexte où la menace terroriste demeure à un niveau élevé. Cependant, le maintien de cette extension particulièrement significative. Au-delà de cet événement n'a plus de raison d'être. Dans le cas contraire, se poserait directement à nous, la question de la proportionnalité de de la mesure. Enfin, les enquêtes administratives seront effectuées par le Service national des enquêtes administratives et de sécurité. La, les, l'élargissement du Champ de l'application de l'article L 211 tirer 11 tirer hein du CSI va nécessairement entraîner une charge de travail supplémentaire. Pour le S N. AS dépendant de la DGPN le dimensionnement de cet organisme en termes de personnel sera-t-il assuré le nombre d'outils informatiques supplémentaires nécessaires à l'application de ce niveau dispositif est-il évaluer, compte tenu de ces considérations, nous vous proposons de limiter dans le temps. L'ex et l'extension exceptionnelle de la procédure de criblage envisagée par ce projet de loi. Si monsieur Chantrel madame la rapporteure avis sur le 65 et le 28. Merci. Madame la présidente. Alors, nous comprenons. L'enjeu de ces deux amendements qui visent à réduire. Le Champ de l'extension de la procédure de criblage telle que prévue par le texte. Ah, effectivement, nous avons aussi des inquiétudes que nous avons émise sur la capacité du cinéaste, a assuré le le le le criblage de toutes ces personnes supplémentaires notamment les participants et ceux qui seront dans les fan-zones. nous ne pensons pas que vos amendements soient les bonnes solutions notamment sur l'amendement 65 de monsieur Besnard Roche qui vise à limiter la procédure pour les participants donc extraire les participants de cette mais en même temps vous supprimez l'obligation d'avis conforme de l'autorité administrative, ce qui rend le dispositif inconstitutionnelle et donc c'est pour la raison pour laquelle nous donnerons un avis défavorable. Quant à l'amendement numéro 28 de monsieur Chantrel, il vise lui a limité la procédure de criblage uniquement aux Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby. Nous pensons, nous au contraire qu'il doit être pérennisé, parce qu'il y aura d'autres grands événements après comme les Mondiaux de cyclisme pour lesquels cette procédure sera utile à la sécurisation donc ce sera aussi un, un, un, un avis défavorable. Merci madame la rapporteure. Monsieur le Ministre même avis sur les deux amendements. je mais. Il n'y a pas de demande d'explications de vote, je mets aux voix l'amendement 65 qui a reçu 2 avis défavorables. Qui est pour. Qui es contre. Qui s'abstient n'est pas adopté, je mets aux voix le l'amendement 28 qui a reçu 2 avis défavorables qui. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté. Je me vois l'article 10 qui est pour. Et contre c'est il est adopté. À l'article 11 amendement. Monsieur Folliot, demande la parole sur l'article. Monsieur Folliot. merci madame la présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bien entendu, au niveau de notre groupe et puis demande ce qui me concerne, tout au moins je voterai ce texte vous dire hein. Un point est un élément qui me paraît important, essentiel puisque. Si ce texte. Fait référence aux Jeux olympiques. Cela a été dit à plusieurs reprises il y a d'autres événements qui vont précéder les Jeux olympiques, notamment la Coupe du monde de rugby. Donc en 2023, qui est un élément important et est essentiel et qui est cher à notre coeur pour nombre d'entre nous et pour la totalité d'entre nous et avec d'autres événements qui suivront et pour lesquels aussi toutes les mesures que nous allons prendre parce que ces enjeux de sécurité sont des enjeux importants et essentiels donc vont permettre de pouvoir expérimenter. Donc avant. Au titre de France 2023. Donc les mesures qui seront proposées dans le cadre de ce texte de loi mais aussi qui vont nous permettre d'acquérir une certaine expérience pour la suite. Tout à l'heure madame la rapporteure. Vous avez fait allusion aux Mondiaux de cyclisme, qui vont suivre, mais je rajoute entre éléments et un autre événement que nous nous nous espérons que nous appelons de nos voeux. Qui est madame la ministre, la Coupe du monde de rugby à XIII, donc France 2025 qui sera aussi un événement important et et pour lequel. Je crois qu'il est important de le marquer de le souligner parce que c'est aussi. Un événement qui va concerner nos territoires, avec des enjeux qui seront des enjeux spécifiques en matière d'attractivité. Et en matière aussi d'inclusion puisqu'il y aura 4 événements en même temps la Coupe du monde masculine féminine. Handisport. Et la Coupe du monde pour les jeunes et donc je crois que ceci est important d'être dit d'être souligné. Si cher collègue. Alors, nous passons à l'examen de l'amendement 50. Présenté par Madame Assassi madame la présidente. Merci madame la présidente. Donc cet amendement vise à supprimer l'article 11 du projet de loi. Qui permet donc l'utilisation des scanners à ondes millimétriques à l'entrée des enceintes accueillant des manifestations sportives. Mais aussi pour celui des enceintes accueillant des manifestations récréative ou. Culturelle dans le rapport de notre commission de lois, des lois, je note que cette disposition ne semble pas avoir été demandée par les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques ou les autorités en charge dans la série nous considérons que, bien que des garanties existent, elles ne seront pas suffisantes la mise en place d'un tel procédé est de nature à porter selon nous une atteinte disproportionnée à la vie privée et à l'intimité des participants à ces différents événements. Merci cher collègue madame la rapporteure. Vous avez la parole. corporels à ondes millimétriques. Sont utiles. D'autant qu'ils seront installés à la demande des organisateurs. Et donc, ça laisse la liberté, c'est un outil supplémentaire donc avis défavorable. Si Monsieur le Ministre. merci ma la présidente peut-être quelques instants madame la la sénatrice pour cette question très intéressante des scanners à ondes millimétriques parce que ceux qui nous écoutent doivent se dire sans doute que c'est un appareil un peu étonnant et pourrait faire croire par votre amendement de suppression qu'il s'agit de quelque chose d'exorbitant du droit commun. D'abord ils existent ces scanners à ondes millimétriques et ils sont dans nos aéroports parisiens pardon Madame Assassi excusez-moi. Désolé. Et donc ils existent dans les aéroports parisiens. nous nous empruntons ces aéroports parisiens nous passons. Dans ces scanners à ondes millimétriques. Quand est-ce qu'ils ont été installés. Pardon de dire Madame Assassi. Dans le gouvernement d'avance ce gouvernement-ci

qu'un prix, un ordinateur cascadeurs. Surtout en ce qu'il respecte les règles que nous imposons aux ondes millimétriques, c'est-à-dire que la difficulté des scanners à ondes millimétriques c'est il peut constater un certain nombre de choses qui relèvent de la vie personnelle des opérations des des des formations des des handicaps et ce que nous imposons aux aéroports parisiens et ce que nous appellerons donc au scanner millimétrique. Dans le cadre des grands événements sportifs c'est de remplacer. Évidemment ces formes et parfois. Ses incursions dans la vie personnelle qui peut faire naître un certain nombre de débats, je peux tout à fait le comprendre par des carrés et des cubes qui en fait signal selon la couleur et sur la grosseur de ses carrés les cubes, non pas le corps de la personne, mais s'il y a quelque chose de.

comme on n'aura pas la sécurité privée je résume hein il faut ne ne ne pas hésiter à prendre l'armée. Je crois qu'avant d'arriver à l'armée, qui est une me semble-t-il la dernière la dernière chose que peut faire le gouvernement ne sont pas tellement fait pour faire des palpations de sécurité me semble-t-il, je devrais d'ailleurs souligné qu'avec la ministre des Sports et aussi la question de la féminisation de la sécurité privée, c'est un autre un autre sujet pour pouvoir. Et vous éventuellement répondre à l'afflux de ces personnes. Bien ce qui se présente dans les lieux. Contrôlés par ces scanners millimétrique au moins le scanner permet de passer tout le monde sans distinction de genre, ce qui peut raison résout aussi le problème de la question entre femmes et hommes et. Contrôle par des personnes qui se disent ni ni familial. C'est une question qui est évidemment importante pour l'organisateur et et pour les services de sécurité avant d'aller vers l'accès que pourrait donner monsieur Assouline au recours à à l'armée. On a peut-être à certains de nos technologies qui peuvent nous aider à payer ou à compléter la sécurité privée donc je ne voudrais pas que par votre amendement madame la sénatrice pour pour dire on a ce lourd ce que je pense vous puissiez nous encourager à recourir à l'armée parce que ce serait quand même une drôle de démonstration du groupe communiste que demandent mise intérieur de recourir à l'armée pour contrôler les gens la la la, après avoir appris que vous étiez. Défavorable au gouvernement Monsieur Hollande j'aurais donc appris que vous souhaitiez l'armée. Ce qui, évidemment, on ne peut pas être acceptable dans cette assemblée, à cette heure tardive, et même si les communistes ont beaucoup changé. Je crois que là vous allez un peu trop loin, avis défavorable. Alors monsieur Assouline. Vous avez la parole pour explication de vote. Bien comme. En fait j'avais un amendement d'appel après j'ai dit je l'enlève. Et puis malgré ça. Vous avez mis le débat donc l'appel a réussi sans que je le dépose. C'est pas mal. Écoutez. Pas de caricature. En réalité, vous êtes venu un jour nous dire que on pouvait plus faire les festivals culturels parce qu'il y avait pas assez de policiers pour faire tout ça et puis vous nous avez même rajouté que les sociétés de protection et cetera. Ça nécessité beaucoup beaucoup de de de personnel pour ce moment-là et que on était même pas sûr encore aujourd'hui de pouvoir les former parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pas pour surveiller une boîte de nuit ou quoi c'est. Ils doivent avoir. Un pedigree en tous les cas et une formation. De de ce niveau. Donc moi quand on me dit que il y a un tel événement qui va se passer notamment à Paris mais que. Le ministre de l'Intérieur, le chef de la police me dit bah il y a pas assez de policiers. Et en plus la sécurité privée, il y en aura peut-être pas assez. je me dis que il y a. L'armée qui. N'est pas là pour venir avec les tanks et tout ça donc. Ne caricaturez pas bon je je. Qui qui est, qui assure dans ce pays des tâches de protection civile à différents moments exceptionnels. Très. Rassurantes, c'est des hommes. Qui sont au service de l'État et au service de la protection. De nos concitoyens et qui peuvent très bien venir pallier si c'est nécessaire. Donc, c'était ça le sens de mon amendement mais comme certains ont voulu. Mettre autour du mois armée. Quelque chose qui pouvaient effrayer ou être très sécuritaire. Ce qui n'est pas mon engagement ni mes valeurs. Mais je m'attendais pas. Ça vous parce que vous êtes plutôt. Très sécuritaire. Au sens. Non, non, au sens. pas très ouvert du terme. Donc voilà je voulais justifier. Je voulais justifier pourquoi je pense à ça uniquement par efficacité et devant les propos qu'il pouvait désorienter et même. Faire que les citoyens soient inquiets. Donc je l'ai retiré mais j'ai aussi répondu à à ce que vous avez dit. Merci monsieur Assouline. La parole est à monsieur le président Laurent Lafon. Merci monsieur le ministre d'avoir ouvert un débat qui n'était pas dans le texte de loi et en plus que le sénateur Assouline qui, un moment avait été tenté de lancer la l'avait rôti avait retiré son amendement. Donc vous vous posez la question de l'armée et je ne peux pas ne pas intervenir puisque j'avais initié avec un grand nombre de membres de la commission de la culture il y a quelques semaines une tribune dans Le Monde. Qui concluait sur le fait que probablement on on recourait à l'armée pour les Jeux olympiques, beaucoup de gens participent, partagent cette idée du reste dans le rapport de la Cour des comptes paru il y a quelques jours c'était écrit aussi noir sur blanc comme une hypothèse qui devenait de plus en plus réaliste et crédible. Compte tenu de la difficulté, même si nous le regrettons. De trouver les 22.023, 1000 personnes nécessaires pour que les sociétés de sécurité privées. Assurent les tâches. Que vous souhaitez leur assigner. Alors ma question, monsieur le ministre, elle est, elle est simple, quand est-ce que le scénario du recours à l'armée sera officiellement annoncée et qu'on pourra enfin dire les choses de manière claire plutôt que de les sous-entendre comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Et ma question est simple, j'ai cru comprendre d'ailleurs à à travers votre intervention tout à l'heure que c'était pas un scénario exclu alors que il y a quelques semaines, vous étiez beaucoup plus réservé sur cette hypothèse du recours à l'armée. Quand est-ce que ce recours sera annoncée ou est-ce que vous nous dites que, définitivement, il n'y aura jamais le recours à l'armée pendant les Jeux olympiques. Si Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. pardon Madame Assassi excusez-moi j'avais pas vu. Vous avez jamais rien. Madame la présidente, j'aimerais bien qu'on en revienne à à mon amendement numéro 5. Et non pas de celui qui a été retiré. En simplement pour dire, Monsieur le Ministre. Bon. Rappeler ici quand même que l'utilisation des scanners Miley millimétrique ont ont été utilisés pour les Coupes du monde de football en Russie

palpation, ce qui n'est évidemment pas la proposition qui est faite. Dans ce texte, voilà encore une des raisons pour lesquelles nous avons demandé la suppression de cet article. Merci madame Assassi Monsieur le Ministre. Pour répondre à la question du président là font et à l'interpellation du du du sénateur a souligné finalement à tous ceux qui s'intéressent à cette question. D'abord je veux dire aux c'est un signe que nous avons supprimé avec la ministre des Sports culture aucun festival. Voilà et aucune épreuve sportive et aucune fête. Régionale local. Nous avons cependant réussi avec les élus locaux avec le festival en expliquant les contraintes de l'État à les décaler. que le Tour de France arrive quelques jours de décalage et à Nice et pas à Paris. En 2024, ça paraît de bonne Intelligence. Je voudrais quand même rappeler ici Monsieur le Sénateur parce que. Ne caricaturez pas non plus mes propos, je voudrais vous dire l'année que nous allons vivre et que va vivre l'aide d'autres pays et donc le ministère de l'Intérieur. Coupe du monde de rugby. Ça a été dit par le sénateur Folio c'est le 5ème événement mondial c'est si nous avions que la Coupe du monde organisée nous serions. Tous pas que sportif événement mondial en général du nombre de spectateurs qui arrive sur dans un pays, nous aurions. Que la Coupe du monde de rugby, ce serait déjà absolument formidable et nous prendrions évidemment beaucoup de temps pour en parler

ce qui pose pour pour autant à ça le souci mise au ministère de l'Intérieur, vous vous l'avouerez, notamment en matière. Dans le public. Puis nous allons, je le dis. En passant organisé l'anniversaire, le 80ème anniversaire du débarquement de Normandie je crois que. La vie fait que tous les chefs d'états. Tous les chefs d'État je viendrai pour dans quelques instants vous inquiétez pas vont venir en Normandie au mois de juin et il y a le débarquement de Provence. Alors comme en Provence 80ème anniversaire ou je crois que le président de la République et c'est bien logique pour tous les soldats venus. D'Afrique et et du Maghreb et d'ailleurs pour venir nous libérer dont mon grand-père, permettez-moi de le dire, ça fait plaisir de dire c'est aussi. Un énorme événement organisé les Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques le 14 juillet qui restera à Paris et d'ailleurs Madame, la maire de Paris avec qui je m'entretiens régulièrement va organiser et c'est bien son droit non seulement de défiler les Champs-Élysées avec qui sera ailleurs sans doute que Champs Élysées. À ce moment-là dans Paris au moment où nous organiserons le début des Jeux Olympiques mais le le Paris-Plage et puis évidemment le feu d'artifice du 14 juillet. Ben il y aura une vie à Paris et c'est bien logique en même temps que la vie des Jeux olympiques en 9 mois, nous avons 5 événements mondiaux a organisé en France, ça c'est le 1er point donc je voudrais revenir sur l'épisode qui est désormais passé monsieur le président de la commission mais pour le sénateur Assouline nous n'avons annulé. C'est une prouesse. C'est une prouesse aucun festival aucun d'événements sportifs, on a simplement demandé de décaler à quelques jours près et certains l'ont fait Avignon Les Vieilles Charrues par exemple et c'est tant mieux. Se pose donc la question dans ce mouvement énorme d'organisation et notamment d'ordre public avec la crise du terrorisme que nous connaissons à la fois de notre capacité en matière de sécurité, je crois que la loi d'organisation du ministère de l'Intérieur a montré que les moyens étaient de plus en plus au rendez-vous et je remercie la quasi-intégralité. de la Haute Assemblée d'avoir voté la Lopmi qui permettra des mois de juin, d'avoir cette UFM de gendarmerie dès le mois de septembre prochain, 4 unités de CRS supplémentaires. Donc je crois qu'on est arrivé à un moyen pour le ministère de l'Intérieur qui répond à tous les événements et pas simplement aux Jeux olympiques Symbole, si j'ose dire de ces jeux olympiques. Et puis deuxièmement la sécurité privée. Il nous faut 22.000 agents de sécurité privés pour faire les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ils sont par ailleurs sur sollicité par tous les événements que j'évoquais précédemment par la vie sociale de notre pays et par les événements culturels et cetera que que nous connaissons. La question de la sécurité privée et notamment à Paris ou en Île-de-France, qui concentre l'essentiel bien évidemment des. Épisodes des Jeux olympiques et paralympiques se pose d'une manière, hommes et femmes à recruter. Mais se pose aussi en hébergement par exemple il va falloir que nous hébergeons à Paris et dans sa proche banlieue. 35 à 40.000 policiers et gendarmes. Et. Quelques milliers d'agents de sécurité privés qui ne serait pas parisien. Et avouez que la plupart des agents de sécurité privés que nous connaissons n'habite pas Paris intra-muros ce ce n'pas faire insulte. Ni à Paris ni aux agents de sécurité privée que de le dire, donc il y a d'abord un effet d'hébergement. Donc avant de répondre à la question de savoir combien on a d'agents de sécurité privée. Il faut qu'on résolve la question de l'hébergement et l'hébergement qui connaît des concurrence concurrence hôtelière biologique une concurrence que chacun connaît désormais de personnes qui louent un certain nombre d'habitations une concurrence je mets des guillemets de personnes demandeurs d'asile par exemple que nous logeons à Paris et en Île-de-France qui présentent 50% la demande d'asile national hein c'est c'est un point très important et puis une concurrence évidemment des agents des forces de l'ordre et de toutes les personnes qui viendront à Paris pendant ces Jeux. Donc d'abord c'est pas tellement une question d'hommes et de femmes, c'est une question, où est-ce qu'on les loge. Donc ça c'est un 1er problème très important sur lequel nous travaillons bien évidemment, nous sommes à un an de la cérémonie d'ouverture, mais un peu plus d'un an on encore un petit peu le temps pour cela. Deuxièmement le COJO et l'organisateur. Des Jeux olympiques et à se disent, c'est lui qui a lancé les appels d'offres pour les agents de sécurité privés. Il va commencer rend publique une partie des appels d'offres, enfin les dépouiller si j'ose dire qu'au début du mois prochain donc au début du mois prochain nous connaîtrons un petit peu plus des lots fructueux infructueux de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais on s'y prend quand même assez tôt avec Tony Estanguet avec le COJO avec la ministre des Sports, ici présent, pour pouvoir rattraper un certain nombre. De l'eau qui serait pas fructueux. Soit parce qu'on va effectivement travailler à ce que tous les gens qui ont une carte de Sécurité Privée puisse pro-prendre ce travail, on a créé dans la loi sécurité globale une carte spécifique. Monsieur le rapporteur Hervé sur les grands événements qui va commencer à couvrir ses effets dans quelques semaines, quelques mois, on a changé l'intégralité de l'information, le CNAPS, les exigences qu'on demande la sécurité privée et il y a bien d'autres sujets évidemment encore à chercher les étudiants. Les personnes intérimaires et puis toute personne qui va découvrir ou qui vont découvrir qu'il y a des grands événements et qui vont donc participer notamment par la sécurité privée à se termine aujourd'hui sur 22.000 agents de sécurité privés. nous avons à peu près 11 à 12.000 personnes, dont nous savons qu'ils répondent à ses exigences. Donc nous avons bien avancé par rapport à ce que j'ai présenté avec la ministre des Sports dans votre commission. Il y a les personnes et l'hébergement. Et le prix que mettra le COJO pour avoir. Ces personnes bien nous avons constaté direct le Ministre du sauf ce qu'on a pu augmenter de 7% le salaire des personnes qui sont agents de sécurité. Oui parce que c'est quand même des métiers où on n'est pas très bien payés et peu féminisé, donc on a 2 sujets, l'attractivité et la féminisation. Je répondais à Madame Assassi pour son un moment que ça court ça pouvait résoudre la technologie une partie des difficultés pas toutes mais une partie des difficultés en prenant les ondes millimétriques les scanners. On va gagner on palpation. Si je veux dire entendent palpation. Voilà ça c'est un 1er. Ça c'est un 1er point donc ça dépendra des moyens technologiques que nous donne le Parlement et de ce qu'on pourra installer bien évidemment. Ça dépendra aussi de la ville de Paris, monsieur le sénateur de Paris, vous n'écoutez plus mais si Madame Lemaire de Paris obtient effectivement l'objectif des 2000 agents de policiers municipaux. On a besoin de moi, j'en privé et je peux me poser la question, je peux vous retourner la question est-ce que Paris aura ses 2000 agents de police municipale au mois de de de de juillet prochain et si vous êtes capable de m'le signer, je serai très heureux que vous me le signer, mais avec un heure de Paris. Nous n'en sommes, nous n'en sommes pas tout à fait certain et c'est bien logique, donc il n'y a pas qu'un problème de défaillance potentielle de l'État. Peut être que devront nous faire appel à d'autres personnes dans l'État par défaillance d'autres collectivités. On est là pour travailler les choses en bonne Intelligence, bien évidemment et si à la fin des fins, des enfin des enfin des enfin il manque un certain nombre de personnes nous regardons ce que nous pourrons faire mais nous pensons nous qu'un grand pays comme la France est capable de répondre à cet enjeu de sécurité privée. Je terminerai par dire que aux Jeux de Londres. La société s'est effondré. Une des grandes sociétés s'effondre, trois semaines, trois semaines avant le début des Jeux de Londres et aux Jeux de Tokyo alors qu'il n'y avait pas. De spectateurs à cause du Covid. Il y a eu aussi un défaut de sécurité privée, donc c'est un problème mondial. Par ailleurs, c'est une branche qui est en train évidemment de de se construire. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, monsieur le sénateur, donc je ne suis pas du tout défaitiste avec la ministre des Sports, nous travaillons ardemment avec les la sécurité privée des entreprises, que nous remercions qui doivent voilà encore encore ce matin encore ce midi Madame la Ministre. Et nous reviendrons vers le Parlement à votre demande, si vous le souhaitez, je pense que c'est plutôt vers février mars prochain que ne pourrons en tirer des conclusions. Je voudrais redire devant vous et la mise et sport là dit sans doute dans son discours introductif, les jeux olympiques à Paris, c'est une fois par siècle. Les cérémonies d'ouverture en dehors d'un stade, c'est une fois tous les 3000 parce que ça n'a jamais existé. Nous n'avons jamais dans aucun pays du monde, organisée. À organiser une Coupe du monde de football. Une Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques. D'été en dehors d'un stade ou d'un lieu sportif. C'est la première fois que cela se passera. Donc évidemment un certain nombre de questions se posent. Ça fait désormais plus d'un an j'y travaille quotidiennement avec la ministre. Des Sports et on aura parmi les sujets sécurité privée si vous nous réinvité à votre commission. Monsieur le président, l'occasion peut-être en février mars 2. Tailler les choses, je voudrais dire ici que c'est une responsabilité du COJO de leur comité réaction des Jeux olympiques et que l'État est là pour remplacer si j'ose dire, à 100 de défaillances de sécurité si le COJO d'autres collectivités ne serait pas au rendez vous leurs engagements. Merci, monsieur le Ministre. Alors Monsieur Bonhomme pour explication de vote.

m'étonner et de savoir par quel raisonnement et par quelle logique vous en venez à demander à ce qu'on se prive de d'éléments essentiels que constituent des scanners millimétrique, qui sont utilisés régulièrement par des millions de personnes dans les aéroports et qui quand même. Sensiblement et fortement même alléger le travail de sécurisation, ne serait-ce que parce que les scanners millimétré sont quand même essentiel pour détecter les armes pour détecter la drogue et surtout pour éviter la fouille corporelle. Donc je je je ne compte prendre toujours pas enfin si je la comprends la logique. De de notre collègue mais je ne vois mal comment ça vient en ligne avec les objectifs de sécurité qui sont premiers de leur gestion d'événements et de manifestations qui va se dérouler et dans les enceintes et à l'extérieur parce que ont caractère récréatif ou de loisirs. Merci cher collègue. Il n'y a plus de demandes d'explications de vote. Je vais donc pouvoir mettre aux voix l'amendement 50 qui a reçu 2 avis défavorables qui est pour. Qui est contre. S'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 64, monsieur Roche. Si madame la présidente. En fait c'est une modification sur l'alinéa 4 de cet article. Qui vise en fait. À préciser les modalités de recueil de consentement des personnes soumises à l'utilisation de scanners à Orly millimétrique à l'entrée des enceintes sportives. L'inspection filtrage, vous le savez. Ce n'est pas remis en cause ne peut être réalisé qu'avec le consentement des personnes concernées mais les modalités d'obtention de ce consentement ça ne sont pas suffisamment. Après 6h l'espèce il s'agit donc juste de suivre la recommandation de de la CNIL de son avis du 8 décembre 2000 va de à savoir à ce que les informations sur le consentement soit réalisée par voie d'affichage et de préciser que le recueil du consentement relève de la responsabilité des agents chargés de la mise en oeuvre du Kader corporelle ce ça va de Pair avec la la mise en place de l'article rose. Je ne pense pas que ça ça introduise eu de dossiers ont restrictive importante mais par contre ça respecte ce qui devrait être le cas, ceux qui sont les préconisations de la CNIL, Qui peuvent être soumises doit être également réformer qu'il existe un autre système d'un dispositif de contrôle. Hé ben en l'occurrence la fouille pas palpation. Manuelle de telle façon à ce qu'elle puisse en toute connaissance de cause. C'est un choix entre les deux méthodes. Si cher collègue Madame le rapport. Merci madame la présidente. Ce sera un avis défavorable. En effet ces précisions que vous voulez apporter sont d'ordre organisationnel et donc de niveau rédactionnel les scanners corporels à ondes millimétriques. Sont des traitements de données personnelles sont donc soumis à au RGPD qui prévoit la nécessité d'information il appartiendra donc à l'organisateur de prévoir l'information des personnes et de s'assurer qu'ils ont bien émis. Un consentement réel et d'autant que la commission des lois à renforcer l'obligation d'information de l'existence de ce, de, de contrôle alternatifs. Merci. Même avis. Je vous remercie je pas d'explication de vote je mets aux voix l'amendement 64 qui a reçu 2 avis défavorables. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 29 et présenté par Monsieur figurent à l'article L. 613 tiré 3 du code de la sécurité intérieure à l'usage des scanners corporels. La commission des lois et nous le remercions a accepté de retenir le caractère Express du consentement là d'ailleurs apporté d'autres garanties complémentaires. Nous vous proposons de faire le. De même, la même chose en cas de palpations de sécurité de la personne qui refuse de passer par un scanners corporels et nous proposons que ces palpation manuelle puisse être assuré par un agent du même sexe, alors on nous dira que cette exigence est satisfaite. Mais ce n'est pas expressément prévu dans le cas du recours à ce nouveau dispositif de sécurité. Si cher collègue Madame la rapporteure. Vivement avis défavorable. Monsieur Durand a déjà fait l'explication c'est satisfait. C'est une précision inutile prévue à l'article L. 613 3 du code de la sécurité intérieure. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 29 qui a reçu 2 avis défavorables pied pour qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je mets aux voix l'article 11 qui est pour. Qui est contre s'abstient il est adopté après l'article 11 2 amendements identiques. Monsieur bas qui va présenter le.

Monsieur le Ministre Madame rapporteur sur collègue. Il s'agit d'un amendement de notre collègue Françoise Dumont. Chaque année les compagnies de CRS de maîtres nageurs sauveteurs sont déployés sur les communes littorales pour accompagner l'augmentation de la population de touristes se rendant en vacances à la mer. Ces policiers viennent renforcer les effectifs locaux et ainsi permettre le maintien de l'ordre dans les communes concernées pour la saison estivale. Monsieur le Ministre, vous nous avez indiqué que durant la période des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Aucune compagnie de CRS MNS ne MNS ne sera affecté sur les plages françaises elles seront entièrement mobilisés pour assurer la sécurité des sites olympiques. La sécurité des communes littorales sera donc particulièrement difficile à mettre en oeuvre à l'été 2024 mais déjà beaucoup d'élus s'inquiètent que cette disposition puisse se pérenniser les années suivantes. Il convient donc de borner le temps de mobilisation de ses policiers à la seule période requise pour le bon déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de Paris pour 2024 et prévoir comme le propose le 1er amendement qu'à l'issue, ces personnels soient réaffectés sur le modèle habituel dès que possible et au plus tard au 31 décembre 2024. Nous passons à madame De Lattre qui nous présente l'amendement identique 46 rectifié. Merci madame la présidente. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre. C'est un amendement que j'avais déposé en en commission et c'est un sujet dont je vous parle de façon récurrente ici dans, dans l'hémicycle. La problématique de la sécurisation des des plages en mer mais aussi des plages. Sécurité. De. Des plages de notre littoral. Nous attendons 15 à 20 millions de de touristes à Paris nous attendons quelques millions de touristes français et étrangers sur. Nos plages. Vous disposez de 60 compagnies de CRS qui est composé de de 80. Effectif. Ça fait à peu près 4800 CRS que vous allez réquisitionné effectivement. Pour les Jeux olympiques. Nous avons. Ces dernières années ou en tout cas pour 2024, nous envisagions d'avoir 278. CRS MNS. une goutte d'eau pour les Jeux Olympiques mais d'une importance cruciale pour les communes du littoral, puisque ce sont. Des personnels qui sauve des vies. 411. Baigneurs sauvés. L'an dernier en Gironde. Sont 43 fonctionnaires sur 8 communes. Donc les maires par mon intermédiaire vous demande de maintenir cet effectif sur nos plages girondines a minima et si c'est possible sur tout le littoral, elles sont inquiètes ou au moins d'avoir quelques personnels qui vont encadrer les jeunes MNS qu'il va falloir recruter et ça ne sera pas chose facile. Nous n'en avons pas tant que ça. Sinon, pouvez-vous nous garantir que ses effectifs vont revenir dès 2025 parce qu'ils ont une crainte, nous voyons les effectifs baisser d'année en année, ils ont une crainte, que ce soit la dernière échéance donné pour ses effectifs. Pouvez-vous m'assurer que ils seront de retour en en 2025 avec un plan triennal, merci. Si madame la présidente. Madame la rapporteure avis de la commission sur ces amendements identiques. Oui merci madame la présidente alors élue moi aussi d'une commune littorale mais dont les plages sont certainement beaucoup moins attractive que celle de la Gironde. Parce que l'eau, il est plus froide. Néanmoins, nous savons bien que cette question de la sécurisation des plages est un enjeu essentiel pour les mères. Et non, notamment pour l'attractivité touristique. De leur territoire. Et donc nous avons eu tout à l'heure, effectivement le débat aussi parce qu'il y a des inquiétudes sur les autres manifestations qui se dérouleront concomitamment à l'organisation des Jeux olympiques de 2024. C'était sur les manifestations culturelles tout à l'heure, on voit bien que là il y a aussi. Un enjeu et des craintes et des inquiétudes sur cette question de la sécurisation des plages. Néanmoins, il va être intéressant d'entendre le ministre de l'Intérieur. S'exprimer sur ce cette question et rassurer. Les élus locaux

Il fait 32 en Polynésie. Oui madame la sénatrice, évidemment. On a lu beaucoup hésité entre les épreuves de Surf à à Bray-Dunes mais c'était la plage et puis la Polynésie mais bon finalement on a eu pitié la la Polynésie française évidemment sera très heureux de faire les Jeux olympiques en Polynésie dans ce magnifique territoire de la République. C'est triste. Sur les effectifs de police. Et de gendarmerie que nous allons affectés spécifiquement pour les Jeux olympiques à Paris bien sûr. En Île-de-France, évidemment et dans les lieux qui accueillent des épreuves sportives dans des territoires. Parfois, qui vont être très sollicités je pense à Chatou par exemple où il y aura des épreuves très importantes qui vont s'y dérouler. Je le dis pour madame. La sénatrice Bénureau. Le ministère de l'intérieur je pense l'avoir évoqué la commission qui avait présidé Monsieur Buffet et monsieur Lafond réfléchi et maintenant on ne réfléchit plus a agi selon 3 types. D'action. La première, c'est la fin des zones police, gendarmerie de façon temporaire pendant ces épreuves de Jeux olympiques et Jeux paralympiques et de réfléchir non plus en zone spatiale mais en mission par exemple c'est un exemple je ne sais pas d'annonce ici mais prenons Châteauroux. Nous pourrions tout à fait imaginer que les épreuves. Spécifiques des Jeux olympiques soient tenus par la gendarmerie nationale. Et que les axes de transports et la sécurité pour lutter con, la délinquance a tenu par la police. Pendant, Saint-Denis pour imaginer que les transports soient tenus par la police nationale, la gare de Denis et que. La tenue du la piscine olympique par exemple sa tenue par la gendarmerie, un chef, une mission un territoire alors que c'est une commune qui d'habitude est en zone police en zone gendarmerie. J'ai pris ces 2 exemples, ce ne sont pas des annonces, on aura l'occasion de le faire au moment voulu évidemment au lendemain des Jeux olympiques et paralympiques tout le monde on trouvera ses petits Denis sera en zone police et ceux qui sont en zone gendarmerie resteront en zone gendarmerie. Mais vous comprenez bien ce que j'essaie de faire. Monsieur le sénateur. 2ème. Sujet, nous allons affecter aussi structurellement des effectifs de police ou de gendarmerie en plus dans des territoires par exemple à Paris pour la préfecture de police, il y aura une augmentation sans précédent d'effectifs. Rien que dans les 2023. Début d'année le 24. Ces 1000 policiers en plus en plus une année dont 300 d'ailleurs en plus dans les services de transport et des unités de forces mobiles qui feront à demeure de la lutte contre la délinquance à Paris, c'est un héritage pour Paris. Jamais il n'y aura autant de policiers à Paris, pendant et après les Jeux olympiques, je les laisserai à Paris qui structurellement depuis au moins 40 ans manque. De policiers Paris mais je l'ai toujours dit, Paris c'est 40% enfin à Paris et la première couronne parisienne la zone de l'APP, c'est 40% des violences dans les transports en commun de toute la France et c'est un quart de la délinquance de toute la France et c'est tout à fait vrai qu'il manquent structurellement des policiers à Paris et dans les 3 départements de petite couronne c'est un héritage. Donc cela non, ils ne reviendront pas. Mais chacun le comprend, je l'aurais fait si j'ose dire, quoi qu'il arrive je l'accélère parce que les Jeux olympiques et paralympiques et ensuite il y a tous les policiers, les gendarmes qu'on va quelques mois durant. Effectivement. À Paris, en petite couronne, ou dans des. Lieux par exemple à Lille, à Lyon ou à Châteauroux, qui évidemment, si jamais ce n'était pas leur affectation d'origine retourneront, bien évidemment. Monsieur le sénateur, l'affectation d'origine donc, nonobstant l'explication que j'ai eu sur l'augmentation structurelle des policiers à Paris, que nous aurions dû faire, je veux bien donner un avis favorable à votre amendement pour rassurer les policiers, les gendarmes si c'était pas le cas déjà et pour leur dire qu'effectivement, je comprends tout à fait votre demande que, une fois les événements olympiques et paralympiques terminé chacun retournera dans sa chacunière et viendront évidemment renforcer les effectifs. De vos circonscriptions. Respectives. Les zones d'ailleurs Monsieur le Sénateur, je veux ici le dire c'est pas que pour les lieux olympiques par exemple on peut imaginer qu'un département comme le Calvados là encore c'est un exemple, je ne fais pas d'annonce mais c'est un exemple que je peux vous donner, il y a quelques zones police à part quand qui sont plus petites. On pourrait imaginer que pendant un temps où on envoie les policiers soient renforcées qu'quand soit à venir en Île-de-France et là encore il faudra qu'on en discute avec eux dans l'action syndicale avec les policiers, ce soit la gendarmerie qui le temps des trois mois prennent l'intégralité. Des zones, on pense évidemment aux zones côtières par exemple ou à la zone à la zone de Lisieux par exemple et après les Jeux paralympiques reviendront évidemment en zone police, puisqu'il n'y aura pas d'annonce faite, je ne suis pas pour l'échange. Changement de zone. Encore une fois je répète pour parler dans la presse locale de demain, ce ne sont pas des annonces, ni pour le Calvados. Ni pour ça ni. Ni pour ni pour Château pour répondre à la question Madame de sur les CRS, maîtres nageurs ben la sénatrice, vous le savez j'ai été mis ce qui les a rétablis, donc si depuis 2 ans il y a des CRS, maîtres nageurs dans les plages de France, que d'ailleurs je le dis en sans aucune. Provocation vis-à-vis des représentants des collectivités locales et ayant été maire moi-même. Que l'État mais de façon tout à fait. J'allais dire à disposition des communes sans leur demander quoi que ce soit, c'est très important pour ces restes de le faire parce que c'est un, un autre rapport police-population et c'est très important pour. Les communes balnéaires comme les vôtres qui ont besoin d'un renforcement de de présence policière. J'ai dit qu'en 2023 j'ai écrit à tous les maires évidemment nous les, nous les maintenant je les ai même renforcé. Il y avait une augmentation d'effectifs. Sur les plages et ils seront évidemment de retour en 2025. En 2024, je ne peux pas en en conscience et encore une fois c'est une fois par siècle, une fois tous les 3000 ans, je ne peux pas prendre des gens dont la spécialité est l'ordre public, c'est-à-dire d'organiser des grands événements. Mettre des CRS même 300 400 500 ou 600 sur les plages de France. Je pense que Madame la il faut bien comprendre que c'est pas un jeu à somme nulle. J'ai essayé de vous démontrer que Coupe du monde de rugby jusqu'à, je pars à pique pendant un an les CRS et gendarmes mobiles seront sursollicité quasiment pas de jours de congé, il faut qu'il va leur famille il faut qu'il se repose. Faut qu'il faisait des cours de de formation évidemment et on ne peut pas me semble-t-il, oublié qu'en Outre-mer il y a énormément d'utilisation de gendarmes mobiles et peut-être demain de CRS. En Guyane en Martinique aux Antilles en Nouvelle-Calédonie qui va connaître des moments peut-être un peu. Voilà en tout cas il faut faire attention en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie on va devoir envoyer des IUFM, sans doute pour l'épreuve de Surf et puis les élections arrivent bientôt madame. La sénatrice évidemment à Mayotte. Où, évidemment, vous connaissez la situation de sécurité donc il faut pas penser somme nulle métropole. Il faut évidemment la pensée. Évidemment avec l'outre-mer et vraiment je crois que ce serait mal utiliser les policiers, les gendarmes que de dire que ceux qui sont spécialisés dans l'Ordre public ne font pas de l'ordre public et les CRS des plages, ils font un boulot très important mais ils ne font pas de l'ordre public. Ce que j'ai dit aux élus, c'est que je vous ai prévenu un an et demi avant. On a le temps d'imaginer des choses. Et pourquoi pas que des policiers, des gendarmes, je pense aux gendarmes pour PSIG par exemple mais je pourrais penser à d'autres types de policiers puissent faire une partie peut être pas tout mais du travail de présence sur les plages, ce ne seront pas des gendarmes ou des CRS. Mobile. Des gendarmes mobiles et CRS mais ça pourrait être de la Sécurité publique. On peut imaginer des gens de la BAC. On peut imaginer des psys, je vous l'ai dit, qu'ils viennent aider les collectivités locales, c'est vrai qu'en 2024 madame la sénatrice. Il y a commerce va falloir qu'on fasse tout un petit effort. Il s'agit pas de lutter c'est je ai pas que les Jeux olympiques de Paris prennent tout. On va bien partager les choses, je pense que ça on le souci. La ministre des Sports et de moi même mais j'aurai l'occasion de le dire à tous les élus du littoral que j'inviterais d'ailleurs en septembre prochain à Beauvau. Si je suis encore en responsabilité et nous aurons ces discussions franches et on verra comment on peut mettre d'autres dispositifs mais je veux donc donné un avis non positif à votre moment mais par contre, de dire que des 25 évidemment ils seront de retour et je l'écrirai aux maires de France lorsqu'en septembre prochain, on aura passé là. La saison 2023. Alors s'il n'y a plus de demandes de parole. Je vais mettre aux voix les 2 amendements identiques de rectifier terre et 46 rectifié qui ont reçu un avis défavorable de la commission est favorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils sont adoptés. Après l'article 11 toujours, nous avons 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Tout d'abord le 30. Madame Robert le présente. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues par cet amendement. Nous souhaitons alerter le gouvernement sur la préoccupation des élus locaux et des organisateurs des grandes manifestations sportives, récréatives et culturelles au regard des coûts supplémentaires que vont entraîner que va entraîner la sécurisation de leur installation. Le projet de loi comprend en effet de mesures prévoyant le déploiement des caméras augmenter et l'installation des scanners corporels. S'agissant des collectivités locales. Le nouveau dispositif constitué par les caméras augmenter va avoir un impact économique et financier pour les communes qui expérimenteront le coup recours aux traitements envisagés s'agissant des scanners corporels et même si la commission des lois a précisé qu'ils ne pourront pas être imposés aux organisateurs, les coûts d'acquisition et de fonctionnement de ces appareils seront à la charge des gestionnaires d'enceintes accueillant les manifestations sportives, récréatives au culturel qui rassemble plus de 300 spectateurs ils entraîneront ainsi une charge d'amortissement à moyen et long terme, le service d'ordre au sein même du lieu où se déroule la manifestation ainsi que le remboursement à l'état des dépenses supplémentaires occasionnées par l'intervention des forces de police et de gendarmerie aux abords de la mairie station représente déjà des charges considérables. Ni l'exposé des motifs du projet de loi ni son étude d'impact, détaille les conséquences financières consécutives aux nouvelles obligations de sécurité envisagées par ce projet de loi. Dans ces conditions, le gouvernement doit nous dire s'il a estimé à combien s'élève le coût de la sécurisation des jeux et comment il compte accompagner financièrement les collectivités ainsi que les organisateurs intéressés lorsque ces derniers recourront aux caméras augmenter aux scanners corporels. Je vous remercie.

qui va exactement dans le même sens. Il a pour objet de demander en fait une évaluation du coût pour les collectivités territoriales. Représenté par la mise en place de caméras augmenter dans les communes qui procédera donc à l'expérimentation. La Cour des comptes je rajouterai dans ce rapport sur l'organisation des JO et des Jeux par la. Qui a, qu'elle a transmis au Parlement au mois de janvier alerter sur l'équilibre budgétaire de l'organisation des Jeux sur les coups supposés pour les collectivités territoriales. Nous sommes que l'État n'a pas pris en compte l'impact économique pour les communes qui expérimentent le recours à ces nouvelles caméras ni même cet impact d'ailleurs en cas de pérennisation aussi l'étude d'impact du projet de loi n'est pas détaillé. Elle ne permet pas de supposer le coude Real de ce nouveau système et donc nous proposons au gouvernement d'établir un rapport sur le sujet. Merci madame la présidente à leur traditionnellement nous sommes. Défavorables et nous ne rompront pas avec cette habitude aux demandes de rapport sur le premier amendement. c'est une double demande de rapport sur l'article 7, la vidéoprotection intelligente et sur l'article 11. Les scanners corporels. Ce qu'il faut savoir c'est que sur et le 2ème amendement pardon pas clair, ce sera uniquement sur la vidéoprotection intelligente sur la vidéoprotection intelligente il y aura déjà un rapport puisque c'est l'objet de l'expérimentation qui. Mènera un rapport sur l'ensemble de ce dispositif dont les. Enjeux bien évidemment. Globaux sur les les les scanners de vidéoprotection. Nous pensons que ça rentrera aussi dans dans la demande d'amendement de rapport introduite par nos collègues de la commission de la culture auprès de la Cour des comptes sur le coût global et l'organisation des Jeux olympiques. avez vos amendements le mérite de poser quand même la question fondamentale des enjeux pour les collectivités locales qui s'inquiète beaucoup sur notamment. Le les coûts, les charges concernant la mise en oeuvre de ces dispositifs donc peut-être que Monsieur le Ministre, pouvoir nous rassurer. Merci madame la rapporteure. Monsieur le Ministre avis du gouvernement. Oui ben je je ne peux nier me le dire que Madame la rapporteure. La Cour des comptes suit évidemment extrêmement. À l'euro près le fonctionnement du ministère de l'Intérieur dans le cadre des comptes de. L'organisation générale des Jeux olympiques d'ailleurs le ministère de l'Intérieur, vous l'avez voté d'ailleurs je me semble-t-il dans la Lopmi, j'en suis même certain. Les 200 millions d'euros de crédits spécifiques du ministère de l'intérieur qui concerne. La sécurité des Jeux olympiques. Donc je crois que nous avons tout ce qu'il faut, si j'ose dire dans le rende compte le rendu compte puisque d'abord, on est à disposition évidemment des des commissions mais nous devons chaque année et notamment à la fin de l'exercice budgétaire 2024 et 2023 2024 évoquer tous les sujets qui qui nous concerne. Donc je ne vois pas en quoi les rapports nous améliorerait évidemment sur cette information. Mais si vous avez des questions particulières qu'on avait habitude je serais à votre disposition, comme l'a dit Madame la sénatrice concernant d'ailleurs les utilisations de de des algorithmes. Là il s'agit en plus pour une partie d'entre eux de dépensés par les collectivités locales puisque ce sont évidemment des caméras de protection sauf la préfecture de police qui visant particulièrement concernées qui relèvent des collectivités locales, mais même la dépend en partie du budget de la ville de Paris pour des raisons ancienne que certains d'entre vous connaissent bien, donc avis défavorable. Merci monsieur le ministre. Madame de La Gontrie. Explications de vote. C'est des précisions sur. Le mode de financement et donc de facturation de ses services. Pourquoi l'article 7 a donc instaurer un nouveau. Dispositif de sécurité qui s'applique certes aux Jeux Olympiques, vous avez parlé des Budgets de la du ministère de l'Intérieur mais aussi aux manifestations culturelles ou récréatives à partir de là, les collectivités locales organisatrices ou les organisateurs de spectacles. Ont effectivement manifesté leur inquiétude face à une nouvelle norme qui pourrait leur être imposé de mise en sécurité, leurs événements et qui sous-tendrait l'autorisation préfectorale par exemple de telle ou telle manifestation. Nous avons évoqué ce point lors de nos auditions. Effectuées Effectuées par par la commission. Et donc je crois qu'il est très important que, dans cet hémicycle le gouvernement disent précisément si. Ces dispositions sécuritaires. Pourront ou non être imposé par le préfet avant autorisation d'une manifestation culturelle. Que ce soit par une association ou par une collectivité et en toute hypothèse qui en aura la charge financièrement. L'article 40 nous a amené à devoir. Utiliser le détour du rapport. Si nous avions pu nous passer de l'article 40 nous aurions clairement affirmé la notion de charge. Voilà donc c'est très important le monde culturel et les collectivités sont inquiète sur ce point. Merci cher collègue. S'il n'y a plus à Monsieur Bénard, je demande la parole. Oui merci je voulais appuyer précisément ce que vient de dire ma collègue Madame de La Gontrie. Pour la voir en audition mais aussi en dehors de l'audition de la commission des lois pour en avoir parlé et pour avoir reçu beaucoup de. De de mode ou de questionnement à la fois des collectivités territoriales. C'est le cas de chacun d'entre nous je le pense mais aussi d'organisateurs de manifestations culturelles et récréatives, puisque c'est un milieu dans lequel j'ai été pendant longtemps. Je sais qu'il y a un réel souci à ce sujet-là en fait. Pour bien comprendre, c'est exactement ce que vient de dire Madame de La Gautry. Aujourd'hui il y a un certain nombre de. Contrôles supplémentaires dans ton Post qu'ils vont s'appliquer en dehors des Jeux olympiques parce que le texte de loi et bâti de cette façon-là dans ton pas ce qu'il risque de devenir pérenne et dans certains se disent s'il devait être pérenne et en dehors des Jeux olympiques pour d'autres manifestations à un moment donné on peut nous demander de de d'avoir au de mettre en place ce type de contrôle obligatoirement pour avoir l'autorisation administrative pour organiser un certain nombre de manifestations. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que pendant les Jeux Olympiques bien entendu cela relève du financement de l'État. Mais en dehors des jeux olympiques, monsieur le ministre. Aujourd'hui la question est posée et donc où souhaitant avoir des éclaircissements.

Personne. N'oblige une collectivité. À avoir des caméras de vidéo protection pour organiser un événement aussi important soit-il. Sinon ça fait très longtemps qu'on n'aurait pas autorisé la braderie de Lille. Ou telle ou telle festivals dans des villes qui n'avait pas assez caméra protection et c'est heures et d'ailleurs si le préfet l'avait fait à l'époque où le ferais il serait évidemment sans doute. Traîner pour abus de pouvoir. Devant le tribunal administratif. Nulle part dans ce texte il est écrit que 2 pourrions conditionner des événements sportifs, culturels culturels en l'occurrence pour madame de La Gontrie évoquée par le fait qu'il ait d'Intelligence artificielle dans telle ou telle caméra. Bon, c'est un moyen supplémentaire, donner à ceux qui sont au courant la compétence des caméras de vidéoprotection qui a la compétence des caméras du du vidéoprotection 3 types de personnes, soit l'État par la préfecture de police point donc oui c'est l'État pour Paris qui paiera l'intégralité des montants que nous mettons sur l'installation des caméras. Vous le savez bien mais en plus de l'Intelligence artificielle qu'on il appliquerait après tout la plupart des sujets s'applique évidemment à Paris. Les collectivités locales, en dehors de Paris. Donc c'est aux collectivités locales de choisir si elles mettent des caméras et si elle souhaite mettre Intelligence artificielle. Dans ces caméras y compris pour les Jeux olympiques et paralympiques. C'est leur compétence c'est donc eux L pardon qui paye l'étape abonder comme on le fait avec les filles pudeur, vous l'avez augmenté ou les multiplier par trois notamment pour l'année olympique pour l'achat de tels ou tels logiciels l'Intelligence artificielle qui s'appliquerait à qui, à ses caméras par exemple la ville de Saint-Denis ne dépend pas de la préfecture de police, nous avons octroyé au maire de Saint-Denis, à sa demande un million d'euros. Un million d'euros. Pour les caméras de vidéoprotection par de Saint-Denis. Si le maire de Saint-Denis, ne voit pas d'inconvénient et souhaite installer l'Intelligence artificielle dans ses caméras et ben nous l'accompagnerons financièrement mais il est évident qu'il prendra une partie de de de la part de cette dépense, je rappelle, bac à Marseille, l'état, le gouvernement du président de la République finance 80% mais dans. Messieurs les élus, vous qui géré des collectivités locales, 80% d'installation de caméras de vidéo pour toute protection. Bon donc il y a des collectivités et puis ensuite il y a on en a parlé rapidement tout à l'heure. Les organismes type RATP. SNCF dont vous avez manifestement accepté par le vote majoritaire de cette Assemblée de les doter d'Intelligence artificielle. Et il leur appartient évidemment d'appliquer ou non l'Intelligence artificielle. Si elle le souhaite, dans des conditions encadrées par le préfet et et qui dépenseront l'argent qui correspond évidemment à la sécurité dans ces transports, nous souhaitons je dis devant le ministre des Transports que et la RATP et la SNCF utilise. Mais. Mais je madame Gontrie vous dites et festivals il n'est nulle part écrit. on nous exigeons quoi que ce soit pour organiser un festival. Voilà c'est ça n'a jamais été le cas encore une fois si cette logique prévalait dans l'État d'abord, je pense que ce serait cassé par le tribunal administratif, bien évidemment. Mais surtout, elle aurait déjà empêché un certain nombre de personnes d'organiser d'énormes festival d'énormes. Rencontres sportives ou festives. Sans qu'il de caméras de vidéoprotection. On l'a jamais exigé de n'importe quelle collectivité y compris celle à qui on disait tous les jours qu'il fallait installer des caméras de vidéoprotection. Je constate d'ailleurs que beaucoup d'élus. Qui auparavant ne souhaitait pas la vidéoprotection désormais des installe voilà et je pense que c'est une très bonne chose. Quand cette encadré comme nous l'avons définie. D'ailleurs je pense que ça répond aux un moment qu'il a déposé, Monsieur Durand sur les algorithmes. Merci monsieur le ministre. Je pense que là. Tout le monde est satisfait. On va pouvoir donc passer au vote sur l'amendement. Qui a reçu 2 avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Et pour. Qui est contre. Sauf si il n'est pas adopté le 67 qui a reçu 2 avis défavorables même vote. Il n'est pas adopté. Nous revenons au cours normal de la discussion des articles et et c'est l'article. Le huit. Avec une parole de madame Jacqueline Eustache-Brinio, chers collègues. Merci madame la présidente. Maillon clé de la chaîne des transports durant les Jeux, les plateformes aéroportuaires parisiennes ont été désignés comme porte d'entrée officielle des Jeux olympiques et paralympiques 2024 par le comité international olympique. Aussi, il convient d'y assurer le meilleur niveau sécurité dit offrir la qualité de service la plus optimale possible. J'avais déposé un amendement cosigné par 60 collègue créer un un article additionnel à l'article 8 visant à mieux garantir la sécurité. Il a été malheureusement déclarée irrecevable. Aussi de la petite 45. Je voudrais revenir. La question de la gestion des bagages suspects et pourtant clé dans la lutte contre la menace terroriste notamment en période de forte influence et tout spécifiquement lors de grands événements internationaux à venir et notamment les Jeux olympiques, plusieurs fois par jour dans les aéroports, les services de l'État sont mobilisés à la détection des bagages. L'identification de leur de leur caractère suspect et leur neutralisation. Autorisé l'intervention des équipes cynotechniques de l'aéroport chargé uniquement de mettre en évidence un risque. Avant de faire appel aux services de déminage seule compétence pour lever le doute sur un bagage suspect aurait permis des gains de fluidité important en aérogare en évitant le recours systématique au service de la sécurité civile. Cela aurait permis de renforcer plus encore la qualité de service rendu au voyageur sans amoindrir la sécurité.

en modifiant le code des transports. Nous souhaitions tout logiquement. Étendre cette possibilité donnée à la RATP, la SNCF aux gestionnaires d'aéroports notamment. Aéroports de Paris qui accueillera un très grand nombre de visiteurs. Je regrette donc qu'il n'ait pas été intégrées au dispositif et je tenais en prenant cette parole à attirer votre attention, madame la Ministre, sur ce point important notamment pour ADP. Merci madame la présidente. Monsieur le président, madame la rapporteure madame la sénatrice, j'en profite pour dire un mot sur la préoccupation importante ce que vous avez soulevée à l'instant. Je pense que les renforcements de dispositifs et notamment l'utilisation de binômes de maître et le chien, y compris dans nos aéroports est très important, comme vous le savez le milieu intérieur vient de nous quitter, il avait porté loi sécurité globale qui permet un certain nombre de dispositifs et notre lecture de la loi sécurité globale, votée en 2021 et que même si le texte pourrait être clarifiées comme je crois c'était votre intention. Nous pouvons avec cette base législative par décret intervenir y compris pour aéroports de Paris, ce décret est d'ailleurs en cours de préparation et ce que je propose c'est que dans la suite de la discussion aussi cela était nécessaire. Au-delà du texte dit loi olympique si nous en avions besoin nous prendrions les dispositions nécessaires, mais l'objectif est partagé. Nous pensons que nous pouvons l'atteindre. Dans le cadre au législatif actuel. Et si cela n'était pas le cas, nous aurions à prendre les dispositions très rapidement pour se faire, mais j'ai eu l'occasion de me rendre encore très récemment sur les plateformes aéroportuaires parisiennes. Nous avons besoin, même s'il y a là aussi des difficultés de recrutement, d'ailleurs. Nous avons besoin de renforcer nos dispositifs cynophile.

Bonsoir Monsieur le Ministre. Juste un petit regret Monsieur le Ministre. Je pense qu'il aurait été intéressant de discuter dans le cadre de de cette discussion. Du problème de transport de substitution du fait de la défaillance de l'État sur ses engagements de livraisons des des lignes de transport sous vous savez c'est un, un sujet très prenant pour les les élus, la la la région parisienne et je regrette qu'on n'ait pas pu en discuter, là il s'agit de de l'article 8.

depuis les véhicules. Et les emprises immobilières de la SNCF et de la RATP. Jusque là c'est clair et dans le texte. Vous, vous ajoutez ou leurs abords immédiats. Les abords immédiats d'une emprise immobilière, je vois ce que c'est mais les abords immédiats d'un véhicule c'est quelque chose de extrêmement large. Ah. Et nous souhaiterions que vous nous vous nous indiquiez parce que là si on lit le texte, on a l'impression que les, les agents de la SNCF et de la RATP ont une compétence territoriale absolu sur l'ensemble de de la de la région parisienne, donc nous aimerions comprendre le sens exact de votre âge ou. Je vous le répète, sur les abords immédiats, notamment des véhicules. Merci Monsieur le Ministre. Reportage. Oui c'est un amendement de suppression d'articles, donc nous émettons un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Pour ne pas prolonger le suspense j'émettrai le même avis que Madame la rapporteure. Mais pour répondre à la question nous avons. Créé il y a maintenant un peu plus de six mois, un centre de coordination opérationnelle sécurité qui a vocation, sous l'autorité du préfet de police a rassemblé les équipes d'un certain nombre d'acteurs qui seront encore plus important au moment des grands événements internationaux, la Coupe du monde de rugby, à l'évidence mais puisque c'est l'objet qui nous intéresse avant tout les Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024. Ce que nous avons constaté, notamment au moment des événements regrettables du Stade de France, c'est qu'il y avait encore un certain nombre de types d'images sur lesquelles pour des raisons, pour être honnête administrativement un peu absurde. Les agents des opérateurs publics de transport RATP SNCF en particulier sont présents dans ce centre opérationnel qui a vocation justement à faire de la coordination ne peuvent pas regarder tous les types d'images et sont censés. Dans la même salle que leurs voisins. Ne pas se préoccuper ou ne pouvoir pas visualiser un certain nombre d'images, de sécurité et donc qu'il nous a semblé nécessaire dans cet article. C'est pour ça que je souhaiterais que on puisse le maintenir c'est élargir la capacité de participation à ces opérations de coordination au sein du Centre de coordination opérationnelle de sécurité sous l'autorité du préfet de police, on ne change pas sa composition. On ne change pas sa mission. On me permet cette facilité qui est me semble-t-il de bon sens, si on veut que ce centre fonctionne notamment au moment des Jeux olympiques. Merci monsieur le ministre, chers collègues, vous avez la parole pour explication de vote. Alors si on a le présente monsieur Ministre pourquoi vous, vous ne l'avez pas écrit comme ça. Parce que là c'est clair. Là j'ai compris de quoi s'agissait. Sincèrement, votre, votre rédaction elle est. Elle est très difficile à comprendre par rapport à l'objectif qui qui lui. Est beaucoup plus clair. Vous avez rajouté un membre de phrase, je pense qu'il aurait fallu rédiger complètement l'article. Merci madame la présidente. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Pardon, madame la présidente, je ne prolongerai pas inutilement et les bas simplement d'un mot, si on peut clarifier la rédaction, je suis tout à fait prêt dans le la navette parlementaire à le regarder mais je voulais être clair sur l'objectif. Alors nous maintenons et nous mettons voix l'amendement. Il est retiré. Je vous remercie. Nous passons 66 Monsieur Bénard Roche. Merci madame la présidente, bonsoir Monsieur le Ministre, vous faire un résumé très succinct en 2 mots. Vous savez on a un petit dada depuis un moment avec certains de mes collègues, c'est qu'en fait on étudie. Un projet de loi sur les jeux olympiques et paralympiques un peu renseigné, on a vu les dates et finalement on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'articles ou on se dit tiens, ça correspond pas, c'est pas les JO c'est pas dans les bonnes dates, donc on se pose des questions vous les pose dans les poste de rapporteur. On essaie d'avoir des réponses on n'y arrive pas toujours, voilà donc c'est un peu le résumé, je vous l'ai fait brièvement puisque vous venez d'arriver. et donc cet cet amendement. En fait c'est ça va dans le même sens parce que l'article 8 telle qu'il est présenté dans le projet de loi il élargit les possibilités de visionnage des agents des services à terre, de la sécurité. Mes collègues viennent de le dire de la SNCF et de la RATP. Voilà, tout ça c'est assez clair aux emprises immobilières aux abords, mais vous allez vous allez éclaircir les abords. Des transports des d'accord voilà par contre en dit. cet abonnement OK surtout si vous l'éclaircissent et mais. Pourquoi le circonscrit pas dans le temps. Pour l'appliquer seulement pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques Vu de l'autre côté de la façon dont on envisage de prétexte pour inscrire des mesures dans droit commun alors qu'elles sont liées à l'organisation de d'événements d'ampleur et qu'elle relève de mesures de sécurité de nature exceptionnelle je rajouterai ça fait la 10ème fois que je les cite, ils vont être contents que la CNIL a révélé que la possibilité offerte à ses agents de visualiser davantage d'images de systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel de doit pas conduire à étant leurs compétences telle que définie par les textes doit leur permettent d'utiliser les images transmises à d'autres fins que celle prévue en l'absence donc de toutes ces garanties de temps et d'utilisation. Il nous semble pertinent de décider ou de marqué dans la loi qu'il ne faut pas pérenniser cette extorsion de visionnage des agents en dehors de la période des Jeux olympiques. Madame la rapporteure. Avis de la commission. dans le temps de ce dispositif et on sait bien que cette coordination de la visite du visionnage des images via le Seco. Est nécessaire pour assurer la sécurisation, en dehors et au-delà. Simplement des Jeux Olympiques, on l'a vu avec. La finale de la Ligue des Champions. Au Stade de France et donc nous pensons que c'est un Nuzzi utile d'autant plus que de nombreuses garanties ont été introduites dans dans le dispositif pour en assurer la constitutionnaliser et on sait que le Conseil constitutionnel est extrêmement vigilante sur ce sujet-là, donc on l'a vraiment bordé. Donc ce sera un avis défavorable. Merci madame la présidente madame la rapporteure. Monsieur le sénateur. Même avis que Madame la rapporteure avec les mêmes raisonnements et les mêmes arguments. Petite hein, j'ai un petit peu suivi les débats enfin intégralement depuis le début de la séance discrètement sur le côté droit de l'hémicycle géographiquement. Mais donc j'ai entendu effectivement remarque dans le même sens, en l'occurrence comme l'a dit Madame la rapporteure. Il nous semble que, même si évidemment cette. Disposition le complément je l'ai dit tout à l'heure, en réponse à monsieur le sénateur, je crois, de bon sens pour que fonctionne bien ce Cecos est lié directement aux Jeux olympiques et paralympiques en effet puisqu'on ne peut pas rater par une mauvaise coordination opérationnelle cet événement, un événement de cette ampleur, je crois que c'est une disposition de bon sens qui est un manque aujourd'hui et qui doit durer au delà de ce grand événement international. C'est pourquoi sur ce. Dispositif précis, nous n'avons en effet pas mis de limite temporelle pour la raison que Madame la rapporteure et que je confirme. Alors merci monsieur. Le ministre du tout d'abord Monsieur dessus puis monsieur Ménard Roche. Oui c'est une petite remarque pour reprendre ce que disait ma collègue. De La Gontrie tout à l'heure on parle le transport. Elle voulait s'exprimer sur une forme de privatisation des transports. Parisiens qui concernerait les JO et au-delà pour reprendre les termes de la rapporteure. Et pourtant on n'a pas pu en débattre ici donc je je je suis perplexe face au à l'explication de vote de madame le rapporteur. Si Monsieur dessus monsieur ben rôle. C'est c'est un peu la même intervention. Je suis surpris par la géométrie variable en fait des décisions qui sont prises quelques fois effectivement on relie ça aux Jeux olympiques, il aurait dit, faut surtout pas parler d'autre chose parce que c'est les JO et puis là, certaines fois on nous dit maintenant finalement c'est la bonne occasion pour changer en fait. L'organisation ou la loi parce que en fait ça s'appliquera après les JO, puisque finalement on peut le faire maintenant, donc en fait on est un peu déboussolé là dedans. Je pense qu'il aurait fallu quand même on a essayé de le faire d'ailleurs là à peu fait en commission. Mais je pense que mon collègue. Thomas Dossus le fera tout à l'heure aussi, je pense qu'il faut vraiment changer le titre de la loi ou alors ça devient la loi elle-même et le cavalier de la loi en fait. Or on sait plus. Merci monsieur Roche madame la rapporteure. Oui, pour répondre à, à nos collègues déjà le périmètre de l'Arctique 45 qui avait été extrêmement définies et on a eu l'occasion, Monsieur le sénateur ben Roche de fixer des contours qui était. Déjà précis mais large eu égard à la diversité des mesures qui sont abordés sont dans ce texte. Je reviens, on est là sur la vidéo protection donc la vidéoprotection. C'est un sujet essentiel, qui est traitée dans le texte on a parlé sur la vidéoprotection intelligente, on en a parlé sur la mise en conformité de la vidéoprotection avec le RGPD à l'article 6, on en parle ici avec le visionnage des images du Cecos, tout ça va dans la même logique sur le traitement des images issues des caméras de vidéoprotection ou situé dans les aéronefs.

Et. À l'article 18. Nous commençons par un amendement 5 honteux. Madame de La Gontrie souhaite une parole sur cet article. Merci madame la présidente. Je vais m'inspirer de l'exemple de notre collègue Eustache-Brinio. Et je vais évoquer ici des amendements que nous aurions voulu voir débattre dans cet hémicycle ont été refusées de l'Arctique 45 Profitant de la présence du ministre des Transports sur un sujet qui donc doit considérer les transports j'imagine évoqué ce point car la position du gouvernement est importante. C'est le sujet, et vous allez voir si vous m'écoutez vous allez voir que c'est le sujet. Nous allons devoir ouvrir au 1er janvier 2025, vous le savez fort bien, Monsieur le Ministre. À la concurrence. Le réseau de bus en Île-de-France donc intra-muros et Île-de-France. Vous avez été saisi par 250 élus d'Île-de-France sur la problématique par rapport aux Jeux olympiques. Que posait cette mise en concurrence. Pourquoi parce que il va y avoir une un morcellement en 12 lots du réseau de transport, il va y avoir des besoins de reprise des équipements de la RATP et donc cela va être un processus très lourd qui va impacter nécessairement dans le calendrier. Le bon déroulement des JO. Je suis avec attention vos déclarations et j'ai bien noté que vous étiez ouvert à un éventuel report si vous été demandé mais j'aimerais que vous puissiez ce soir précisé et je regrette de faire perdre un peu de temps notre collègue que cela impatiente aux 250 élus qui vous ont saisi la question de savoir si oui ou non vous allez faire en sorte que le réseau de transports publics en Île-de-France fonctionne le le mieux possible pendant les JO ou si vous allez maintenir cette date du 1er janvier 2025, qui risque de mettre un certain désordre dans cette organisation. Si cher collègue. Personne. Monsieur le Ministre, vous souhaitez la parole. Oui je je ne voudrais pas éludé ce sujet important même si j'ai conscience que. Les amendements qui vont suivre, qui sont très importants aussi. Donc je voudrais dire un mot sur le fond de la logique qui préside à ces amendements concernant les véhicules pour les personnes à mobilité réduite. Mais je voudrais répondre à Madame, la sénatrice. De La Gontrie, car on parle d'une sujet qui n'est pas directement lié aux Olympiques je tiens à le préciser parce que le sujet c'est de savoir si. Le service public des transports en Île-de-France. Et de là dessus que vous avez interpellé le gouvernement, la Première ministre et moi-même fonctionne bien ou pas. Et cette question se poserait indépendamment des Jeux olympiques et paralympiques. Je vais très synthétique et très claire, je l'espère. Il y a une loi qui a été votée en 2009. Pour l'ouverture à la concurrence progressivement des transports publics dans un cadre européen, pas seulement en Île-de-France France d'ailleurs, mais y compris en Île-de-France. Cette loi date donc il y a 14 ans. Et elle a fait ensuite l'objet d'une discussion avec les autorités européennes puisque tout cela part d'une discussion européenne en 2013. Cette loi et l'accord de 2013 qui ont, vous l'aurez noté, été conclu. À deux moments différents sous de majorité politique différente, n'a jamais été remise en cause. Je vous remercie d'ailleurs madame la sénatrice d'avoir utilisé les mots nous parlons pas de privatisation comme j'ai plus longtemps. Non, parlons d'ouverture à la concurrence qui est fondamentalement différent puisqu'on le fait en cas d'ouverture à concurrence dans la cadre de service public définies par le législateur, voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. En effet, moi je l'ai dit, la concurrence, l'ouverture à la concurrence n'est pas. Une fin en soi, c'est un outil, c'est un moyen et donc le but c'est que le service public des transports en Île-de-France comme ailleurs fonctionne au moment de jeux olympiques et surtout il y a là puisque c'est le législateur qui a fixé la date du 1er janvier 2025. Moi je l'ai dit ce que c'est cela qui incombe à l'État, le gouvernement et surtout le Parlement. Moi je suis ouvert à ce que cette date puisse être décalé pour que la mise en oeuvre sans revenir sur le principe se faire de la meilleure façon possible, ensuite il y a les autorités organisatrices de mobilité, c'est la région et de le France et si tu Île-de-France mobilités donc je respecte cette compétence. Vous l'avez dit, je crois pas trahir sa pensée. Madame la présidente de région Île-de-France mobilités Valérie Pécresse ne souhaite pas un décalage de l'ouverture à la concurrence et je crois ne pas trahir non plus à penser son propos en disant qu'elle souhaite au nom de la région dans les quelques semaines qui viennent faire une évaluation avec la RATP par ses propres services du processus d'ouverture à la concurrence. Ce que j'ai dit c'est que si il apparaissait, et si c'était le diagnostic et la demande de la région et la demande d'un certain nombre d'élus franciliens dont vous avouerez les 12 dont Sur la qualité de ce processus, la capacité à mener à bien, au 1er janvier 2025. Moi comme Ministre des transports au nom de l'état je serai ouvert à ce qu'on ait un calendrier qui soit revue et qui nécessiterait évidemment de repasser devant le Parlement en faisant cette évaluation attendons ce que la région a à dire en tant qu'autorité organisatrice dans les mois qui viennent et ensuite sans remettre en cause le principe je le défends je l'assume, faisons bien marché. Ce processus quitte si cela est nécessaire à ajuster le calendrier et-ce à leur proposer au Parlement, il faut évidemment que cela soit réglé au cours de l'année 2023 puisque, puisque là nous parlons des Jeux olympiques et paralympiques que l'année 2024 ne serait pas tout à fait propice à ces changements qui doivent être éventuellement anticiper. Merci monsieur le ministre. Alors, nous passons à l'amendement 59 et Slovaquie. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'organisation et l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques 2024 doivent pour être un succès, garantir l'accessibilité. De l'ensemble des personnes, notamment les personnes en situation d'handicap. Il est regrettable que le ratio de véhicules taxis adaptés aux personnes en fauteuil roulant ne soit que de 1,7% sur Paris. Soit moins que la moyenne sur l'ensemble du territoire qui elle est à 2,2% de la flotte de taxis accessibles en Île-de-France. N'est que de 200 véhicules pour 62.000 personnes en fauteuil roulant résidant sur ce territoire cet écart démontre le retard en matière d'investissements et d'accompagnement des sociétés de transport pour permettre de garantir le droit à la mobilité des personnes en situation de handicap. Dès lors, l'article 18 semble. Partir d'un constat juste pour une solution qui ne les malheureusement pas en effet en autorisant le préfet de police de Paris a délivré des autorisations de stationnement aux personnes morales directement et non plus aux véhicules. Nous prenons le risque de favoriser les sociétés de type Hubert a bénéficié d'une autorisation globale pour l'ensemble de sa flotte de véhicules alors même que le nombre de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite est extrêmement faible. Nous refusons de favoriser économiquement des entreprises qui ne respecteraient ni le droit fiscal, ni le droit du travail dans notre pays, je vous remercie. En effet nous avons. Amendé cet article 18. Monsieur le Ministre, en commission des lois dans un souci de respect de la constitutionnalité, parce que nous avons considéré que le fait de mettre un seuil. Autour de 10 autorisations de stationnement pour autoriser. L'accès aux taxis à mobilité réduite ou pour les personnes en fauteuil en fauteuil roulant. Poser un problème au regard du principe d'égalité devant la loi, notamment en matière de liberté de commerce. Et d'entreprendre. C'est pour ça que nous avons préféré l'ouvrir, je pense qu'on aura d'autres échanges et que aujourd'hui nous avons. Ouvert à la fois à ceux qui ont une autorisation individuelle depuis 2014, et à ce aux personnes morales qui ont. Plusieurs autorisations et qui existaient antérieurement. Et donc nous pensons que l'enjeu d'accessibilité des Jeux olympiques. Dans le souci aussi d'ouverture. Et d'inclusion est un enjeu tout à fait louable qu'il faut accompagner donc nous sommes favorables à cet article 18 est donc défavorable à sa suppression. Merci, monsieur le Ministre même vie. Même avis je tiens simplement à dire un mot parce que nous parlons d'un sujet extrêmement important, je tiens beaucoup à cet article, c'est pourquoi je suis défavorable à sa suppression. C'est un article que nous avons porté avec la ministre des sports et jeux olympiques et paralympiques parce que nous avons pris, parmi les engagements essentiels de ville hôte et de pays hôte pour ces Jeux olympiques, l'accessibilité pour les Jeux olympiques et comme héritage aussi de ces jeux olympiques et paralympiques et notamment pour Paris et la région parisienne, nous avons pris cet engagement fixé cet objectif 2000 taxis pour les personnes à mobilité réduite, sachant qu'on parle. de deux à 300 sont les estimations au maximum taxi aujourd'hui équipés pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est un changement majeur que nous devons réussir et nous avons pris déjà des dispositifs un décret d'aide à l'équipement des taxis PMR. Il y a déjà quelques mois au printemps, qui pourrait être très franc, ne donne pas les résultats escomptés. Peut être parce que nous avons pris un peu trop de délais pour les procédures de versement de l'aide, mais surtout parce que les taxis individuellement se saisissent encore assez peu de cette aide publique de cette tête de l'État et on ne va pas assez vite et pour être très clair, si on s'en tient là, on n'atteindra pas l'objectif des 1000 taxis prr très loin de là et donc nous avons avec Amélie Oudéa-Castéra voulue et Geneviève Darrieussecq qui liait cet article de la loi olympique parce que c'est un levier supplémentaire. passer par les personnes morales, c'est qui nous vend ses créatif, ça se fait uniquement pour l'équipement de véhicules PMR et pour être très clair, c'est un moyen d'accélérer les commandes de véhicules et il y a urgence et c'est même le dernier délai au moment où nous sommes pour faire ses commandes et qu'il y ait des véhicules équipés et qu'on atteigne l'objectif 2000 taxis prr qui est essentiel dans la réussite de chez eux et de leur héritage alors un point pour être très précis, le périmètre est strict. Merci pour la réécriture qui a permis de le préciser les personnes morales dont on parle ce sont des sociétés de taxis cela ne visera pas dans la rédaction de l'article, vous pouvez le vérifier, je vous en apporte la garantie des sociétés comme uber, ne serait-ce que parce qu'elles ne sont pas basés en France, pour l'heure, c'est au siège social et le rétablissement juridique et qu'elles ne sont non pas si cela vous rassure au dispositif donc oui j'assume d'activer de manière créative avec la ministre avec Geneviève Darrieussecq et si le Sénat et le Parlement, ensuite on est d'accord globalement ce dispositif original pour ce but précis essentiel et pour accélérer avec les garde-fous et les limites que j'ai précisé. l'heure. Retirer le 59 et retirer je vous remercie. Le sang de présenté par Madame la rapporteure Madame Canayer. Oui madame la présidente. Alors c'est un amendement de cohérence rédactionnelle. Que j'introduis sous le contrôle du sénateur mouillé particulièrement engagé sur les questions en faveur des personnes en situation de handicap et ce qu'on vient tout simplement de remplacer la notion de fauteuils roulants pour par celle de mobilité réduite. Merci madame la rapporteure, Monsieur le Ministre. À équiper les véhicules pour les personnes en fauteuil roulant la mobilité réduite. C'est une notion un peu plus large. Honnêtement, je crois qu'on partage l'objectif donc je préférerais que l'amendement soit retiré si vous y tenez, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Alors je mets aux voix l'amendement 100 de de la commission qui a reçu, reçu un avis favorable du gouvernement qui pour. Qui est contre qui s'abstient il être adopté. Je me vois l'article 18 qui et pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Moi ce que je vous propose si vous le souhaitez, c'est de faire. D'examiner l'article 12 puis d'arrêter ensuite si. On va relativement vite, ça nous permet d'arrêter vers minuit et demi. Ou. On s'arrête à minuit. Minuit et demie. Tout le long des. D'accord. Minuit et demie. Allez donc nous revenons au cours normal de la discussion des articles à l'article 12 2 amendements identiques de suppression.

que vous qui le dites, madame la présidente. Nous avons donc à nouveau rapporteur Monsieur Kern. Tout le monde est à sa place, il ne manque personne. Alors on y va. Est assez floue et peu pénalisées de façon forte des situations différentes, par exemple sur la question des billets pour l'entrée dans les stades. Lorsqu'il y a une invitation lorsqu'il y a un billet nominatif. C'est une question mais par exemple on peut avoir un prix de dernière minute et donc on, on voit qu'on pourrait pénaliser la une personne qui se voit prêter ou offrir une place à la dernière minute comme quelqu'un qui escalade. Le stade pour y rentrer de façon frauduleuse. La 2ème chose c'est. Sur la question de l'envahissement du terrain. Là aussi il y a plusieurs situations. Et notamment dans le sport populaire. Que ça soit dans le sport professionnel ou amateur. Le fait qu'à la fin du match, un certain nombre de supporters de familles de jeunes enfants rentrent sur le terrain pour célébrer avec les joueurs ou les joueuses leur victoire. Nous semble que. On puisse les pénaliser d'une forte amende, voire même. D'une peine de prison de six mois nous paraît là aussi excessif et donc. Nous pensons que nous mélangeons tout évidemment il y aura besoin lors de la Coupe du monde et lors des Jeux olympiques et paralympiques de protéger l'ensemble des athlètes mais pas de pénaliser fortement les supporters les supportrices qui seraient amenés. À à fêter la victoire de telle ou telle athlète, nous pensons que nous allons trop loin il y a déjà des sanctions qui sont prévues qui sont déjà assez lourde et donc nous nous proposons pas de rajouter un arsenal. Législatif supplémentaire sur ces questions, je vous remercie. Merci cher collègue. Nous passons la présentation du 61 monsieur mais Merci madame école à la présidente, je donne un avis favorable à l'amendement de monsieur Gay. Et le bien va dans le même sens en fait pour rien vous cacher. En fait il existe déjà des infractions qui sont prévues dans le code pénal pour les faits en question. Voilà et en fait il s'agit d'une aggravation de ces infractions pénales. En prévoyant dès le départ une pour primo délinquants. Une amende de 7500 euros. Ça vise mon collègue l'a très bien dit les supporters alors que par exemple le rapport. Ces incidents survenus au Stade de France a bien révélé que les défaillances étaient imputables à la billetterie au plan de mobilité et des supporters alors que la prise en compte des supporters a été insuffisante et et qu'elle a été gérée uniquement sous un angle de Mathias de. Et donc, ça semble maintenant un peu malaisé. De se servir d'éléments de ce type là pour. Rendre la loi plus. Contraignante et est plus sévère encore. En plus il y a un 2ème élément que je préciserai un autre élément en dehors de sécurité. Vous savez très bien que. Dans un certain nombre. De, d'endroits. Les activistes et en particulier les activistes écologistes. Vont être amenés à commettre un certain nombre d'infractions qui nous semble. Par cette loi. Puisque il est précisé que la fraction sera constituée lorsque les personnes se maintiennent entre guillemets sans motif légitime sur l'aire de compétition du dans cette sportive. Or les intrusions non violente. Dans les enceintes sportives certains modes d'action régulièrement utilisé par des activistes écologistes a fallu mener des actions non violentes de sensibilisation sur l'urgence climatique et ces actions là en fait, elle pourrait être avec l'adoption d'une telle infraction et depuis 10 de 7500 euros d'amende pour chacun d'entre eux. Bon pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu du caractère disproportionné de ses peines. Nous demandons nous aussi la suppression de cet article. Merci cher collègue. Monsieur le rapporteur. Vous avez la parole. Merci madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Ces deux amendements identiques. Sont les premiers d'une série qui vise à contester la nécessité d'adapter notre arsenal juridique pour répondre aux défis qu'représentait d'une part les violences survenues au Stade de France le 28 mai dernier et d'autre part, la multiplication des envahissement d'aires de compétition pour promouvoir des messages à caractère politique sans lien avec les compétitions concernées. notre objectif est de préserver la sécurité la neutralité et la sérénité des compétitions sportives et les dispositions qui ont été. Adopté honte d'ailleurs été pesé avec procure Afin de respecter le principe de proportionnalité des peines et celui de l'individualisation. De précision. Une précise, la première c'est que les billets nominatifs ne sont pas des billets individualisé. Donc que ça ce soit clair et que l'intérêt l'intrusion sur une aire de compétition est différente. Encore que l'envahissement festif le festif n'est pas concerné. Si Monsieur donc avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur. Madame la Ministre à vie du gouvernement. Madame la présidente, messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur. En effet mon appareil un avis défavorable dans la mesure où on a absolument besoin pour notre objectif de mieux lutter contre les violences et les incivilités dans les stades de créer, c'est de nouveau délit. délit danse le devine d'intrusion dans un stade par force ou par fraude qui est à la fois contraires aux règles des stades et qui peut perturber le bon déroulement des compétitions et le délit de pénétrer sur l'aire de jeu sans motif légitime qui a peu déstabiliser des périmètres de sécurité créé aussi un risque d'exposition nos acteurs à des compétitions et des risques et puis troubler l'ensemble de la compétition. Évidemment, ces situations ne couvre pas l'hypothèse que vous avez mentionné monsieur le sénateur d'une famille qui serait simplement joyeuses de retrouver une personne victorieuse sur un terrain dans l'hypothèse où tout ça et de toute façon sous le contrôle du juge. Ça ne vise pas du tout ce type de ce type de comportement donc avis défavorable. Madame la Ministre. Monsieur Gay, vous avez la parole pour. Explications de vote. Merci madame la ministre. Madame la présidente, pardonnez-moi madame la ministre, mes chers collègues. Et une question dont on ne parle pas, madame la ministre en élu avait ma présidente de la Seine, Denis. Une des questions pour prévenir l'intrusion dans les stades. C'est chacun et chacune puisse participer. À la fête et une des questions à laquelle nous nous avons été amenés à à discuter avec Tony Estanguet mais ça serait la même chose avec la Coupe du monde de rugby et même pour beaucoup de matchs de Ligue 1 de Ligue 2 de rugby ou d'autres, c'est que évidemment la fête elle puisse s'ouvrir à toutes et tous. Vous avez une question lors du Stade de France, je ne vais pas une robe noire je connais connaît parfaitement la chose mais oui il y avait plein de gamins qui rêvait de voir la la la la finale de Ligue des champions, plein de gens qui avaient envie de voir Karim Benzéma et de d'autres joueurs. Sauf qu'avec des prix de place à 500 voire plus. C'est impossible pour une majeure partie. De la population de la Seine-Saint-Denis aujourd'hui avoir accès à des compétitions sportives et un des grands enjeux dont devrait débattre. Dans un texte sur sur les Jeux olympiques et paralympiques, c'est l'accessibilité notamment sur le prix des places parce qu'aujourd'hui ce que moi se dérouler et pour la Coupe du monde de rugby ou par exemple les packs sont déjà mis en place mais il faut 1000 euros pour arriver à avoir accès, 1000 euros. Aujourd'hui, quel, quel jeune de nos départements peu maître millions euros sur la table pour aller voir un match Coupe du haut personnes pendant monde en tout cas et si les Jeux olympiques et paralympiques. C'est la même chose, là aussi on se met en difficulté, on met en difficulté nos forces de sécurité. Je ne dis pas que ça règle tout. Mais je dis que ça règle en partie le problème et la dernière chose vous pourrez doubler, tripler, quadrupler les amendes les gens qui ont vraiment envie malheureusement de commettre un délit. Le front et ça ne règle aura rien. Donc la question. Prévention et permettent que ces compétitions soient véritablement populaire. Les Jeux olympiques et paralympiques vont se dérouler dans notre département. J'espère qu'il nous le verrons pas qu'à la télévision, je vous remercie.

Vous inquiétez pas je ne veux pas être très long. Je crois je comprends bien qu'en fait. Essentiellement aussi d'ailleurs pour des raisons de retransmission. Télévisuelle et parce qu'en fait les grands événements se voit dans le monde entier parce qu'ils sont retransmis et sont vu par des millions et des milliards de spectateurs et de téléspectateurs. Je comprends bien qu'on veuille tenir ces événements à l'abri de toute manifestation citoyenne et à l'abri de gens qui pourraient venir fêter un certain nombre de choses mais qu'ils ne le peuvent pas parce que le prix des billets, vous l'avez dit devient. Donc si on veut faire du, du sport ou en tout cas des grandes manifestations sportives, une expression. Élitiste de certains modèles de sport, on va y arriver. on va y arriver. À cette. Interpellation sur l'enjeu d'accessibilité en termes de prix des Jeux olympiques et paralympiques. C'est un enjeu majeur, on lui est extraordinairement attentifs, je voudrais vraiment rappeler à cet égard que 50% des billets aux Jeux olympiques sont à moins de 50 euros et que nous aurons un million de billets à 24 euros et. En plus de ces éléments d'accessibilité auquel on a été encore une fois extraordinairement vigilants. Le président de la République a pris la décision de déployer une billetterie populaire 400.000 billets qui seront offerts à une série de catégories de personnes qui en ont besoin, dont notre jeunesse et je rappelle aussi que le territoire de la Seine. Je l'ai exposé tout à l'heure bénéficient de 80% des investissements, c'est évidemment un territoire absolument prioritaire pour nous, dans cette logique. Merci madame la ministre je mets aux voix les amendements identiques, 51 et 61 ans qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour.

Oui madame la la présidente cet amendement tend à rétablir la rédaction initiale du texte de l'article 12. En la modifiant néanmoins à la marge pour tenir compte de de certaines préoccupations cet amendement préserve en effet la nouvelle obligation voulue par le rapporteur de pénétrer dans une enceinte sportive. Muni d'un titre d'accès. En revanche, nous proposons de revenir sur certaines dispositions le souhaitant supprimer la peine de prison de prison opposable au nouveau délit sanctionnant le fait de pénétrer en récidive en réunion dans une enceinte sportive lors d'une manifestation ou de sa retransmission en public comme d'ailleurs souhaité par le Conseil des têtes dans son avis sur le projet de loi, donc on s'aligne sur la position du Conseil d'État. Nous souhaitons également exclure de l'application des peines dont sont passibles les personnes. Ou agissant en réunion ayant pénétré ou tenter de le faire dans une enceinte sportive ou sur son terrain pendant une compétition celles qui agissent dans le cadre d'une action militante non violente. Nous reviendrons sur ces 2 points dans la défense de nos amendements de de repli de considérant surtout que la rédaction de l'article adopté en commission durcit. Suffisamment la peine qui est envisagée. Je rappelle aussi que le montant de l'amende pour les primo-agissant était plus que doublé. En commission. Enfin nous souhaitons nous aussi tirer tous les enseignements toutes les conséquences des événements regrettables qui sont déroulées au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Mais c'est vrai que. Et je pense que nous l'avons démontré. Nous ne souhaitons pas aller aussi loin que certains le le souhaiterez. Je pense effectivement qu'il y a des nuances entre nous, nous disons ce qui ne concerne que les débordements en question au Stade de France sont plus le fait d'une mauvaise gestion de l'événement par le préfet de police en particulier que l'objet d'infraction à grande échelle de la part du public et je n'oublie pas non plus. Les difficultés liées au plan de circulation. Merci monsieur sac hein. Le 12 est toujours présenté par vous monsieur. Oui merci bon cet amendement de repli tend à supprimer la peine de prison opposable au nouveau délit sanctionnant le fait de pénétrer. En récidive en réunion sur le terrain où se déroule une manifestation sportive là aussi douteux dans compte de l'avis du Conseil d'État. Hein je vous donne simplement la lecture de l'extrait de de cet avis. Je cite il n'y a pas lieu de prévoir une peine d'emprisonnement. En effet, dans l'hypothèse où le comportement dont il s'agit, troublerait la compétition ou porterait atteinte à la sécurité des personnes ou des biens il entrerait dans le Champ de l'article L. 332 tiré 10 du code du sport et serait passible d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende. Et dans le cas vous la pénétration ou le maintien sur l'aire de compétition n'aurait pas de telles conséquences. Une peine de prison serait disproportionné, Pour ce qui nous concerne en cas d'intrusion sans conséquence grave sur l'air d'un stade où se déroule la compétition. Ce que nous regrettons, tout simplement, c'est que le sujet de la sécurité soit dans ce cas-là uniquement abordée sous l'angle de la lourdeur de la sanction. Si Monsieur Lozès que monsieur Chantrel pour le 13. Oui, 13 et 14 même puisque ces deux amendements de repli. Ils tendent à exclure de l'application des peines dont sont passibles, les personnes ayant pénétré ou tenter de le faire dans une enceinte sportive pendant une compétition celles qui agissent dans le cas d'une action militante justement non violente. Exemple de propos d'incitation à la haine ou à la discrimination. Nous avons tous et toutes. En fait en tête et ça a été rappelé par par des collègues et les actions militantes qui se déroule pendant des compétitions sportives telles celles des militants enchaînés au filet de de Roland Garros lors de la demi-finale de 1022, pour alerter sur l'urgence climatique. Donc je ne souhaite pas laisser à la presse. Et si l'appréciation du juge. Le fait de savoir si cette action constitue un motif légitime motif légitime qui n'est prévue d'ailleurs que pour le fait de pénétrer sur l'aire de compétition et qui ne sera pas prise en compte dans le cas d'une intrusion dans l'enceinte sportive dont tu traite justement l'amendement 13. Je suis par ailleurs très étonné. De l'argument qui a été avancée ce matin et qui sera certainement reproduit aujourd'hui par notre rapporteur, que cela ne pouvaient être assimilés à des activités militantes. En vertu duquel la diffusion audiovisuelle doit être coupé dès qu'une intrusion a lieu pendant une compétition. Cet argument répond d'abord à une vision très restrictive du militantisme, dont les actions ne sont pas montés dans le seul but d'être diffusée par les médias. Mais pour alerter de façon générale d'événements d'envergure surtout l'argument opposé par le rapporteur ne répond aucunement un autre souci de préserver une action pacifique militante qui devraient ainsi être exclus d'une application des peines de droit commun ici très lourdes comme ça a été rappelé par mon collègue et encore durci par le rapporteur puisqu'elle concerne désormais les primo-agissant et non plus seulement comme dans le texte initial, les récidivistes ou les personnes agissant en bandes. Si cher collègue monsieur le rapporteur. Avis sur ces amendements. Merci madame la présidente Madame la Ministre. Mes chers collègues. En ce qui concerne l'amendement 11 donc cet amendement vise à revenir sur l'objectif même. De l'article 12. Je vous rappelle que le nouvel article L 332 tiré 10 tirer hein vise à sanctionner les activistes qui. Utilisent les grandes retransmissions sportives afin de 10 fois diffusé un message politique. Merci. L'amendement supprime toute sanction à leur égard et constitue donc un appel à troubler toute manifestation sportive avec les conséquences que l'on peut imaginer sur le déroulement de ces événements. Son adoption reviendrait à mettre en péril des retransmissions des Jeux olympiques et paralympiques compte tenu de la multiplication de ces incursions par ailleurs l'amendement supprime également la peine de prison pour les personnes qui s'introduisent par force ou par fraude dans les enceintes sportives en récidive ou en réunion, ce qui revient à considérer que les incidents survenus au Stade de France ne justifie pas de renforcer. Notre arsenal juridique pour un pas pour empêcher leur réitération l'amendement contredit également l'objectif de la commission de mieux sanctionner les primo-délinquants isolé. Donc c'est un avis défavorable. L'amendement 12 qui est un amendement de repli Devlies là encore à ne pas tirer toutes les conséquences des événements survenus au Stade de France où la vie de nombreux spectateurs a été mise en danger à la fois par des fraudeurs et par des délinquants qui se sont introduits par force dans l'enceinte. Je rappelle qu'aujourd'hui le code du sport sanctionne d'un an de prison. Le fait de s'introduire par force ou par fraude dans une entente sportif sportive en état d'ébriété sans condition de récidive ou de réunion. La peine de 6 mois de prison est donc très mesuré. Elle n'a pas été remises en cause par le Conseil d'État qui s'est prononcé défavorablement sur l'autre circonstance de l'intrusion sur les aires de compétition sans violence. Je rappelle à cet égard que la commission n'a pas rétabli la peine de prison. Dans ce cas. Donc c'est un avis défavorable également. L'amendement 13, comme plusieurs qui précédait donc vise à ne pas sanctionner les actions militantes qui viennent troubler ou interrompre la retransmission des compétitions sportives à des fins politiques. Je rappelle que les diffuseurs audiovisuels sont responsables de la maîtrise de Laurence antennes ils doivent donc coupé la retransmission Dès qu'une intrusion a lieu. Chacun a à l'esprit de ces moments où la compétition est arrêté sans explication des commentateurs qui ne peuvent décrire la situation. Ces intrusions ne peuvent donc en aucun cas être assimilée à des manifestations. Ces actions ne participe à un aucun débat démocratique puisqu'elles ne sont pas diffusés. Avis défavorable et même avis, pour l'amendement 14. Il est également un un avis défavorable sur ces, sur ces quatre amendements dans la mesure où on on veut vraiment essayer de traiter l'ensemble des formes de violence et d'incivilité. Ce que je voulais dire sur les primo-délinquants isolé c'est que c'est pour nous très important d'avoir cet effet dissuasif aussi pour ces personnes-là. Rappeler comme vient le faire le, de le faire. Le sénateur Kern que l'avis du Conseil d'État porté bien sûr la peine d'emprisonnement pour l'entrée dans. Le stade en cas de récidive ou de réunions hein. Cette peine de prison. C'était uniquement dessus que portait son son avis. Et s'agissant de l'action militante. Je crois qu'on on ne regarde pas l'intention. Mais les effets, on a pu voir sur un événement sportifs comme le Tour de France que ses effets pouvait être très dangereux, très perturbateur de ces compétitions, et donc au nom de la tranquillité tranquillité de ces événements et de leur dispositif de sécurité. Nous avons aussi besoin de couvrir ces situations. Si même la ministre alors j'ai 2 demandes d'explications de vote monsieur Chantrel pour commencer. c'est c'est quand même assez problématique. Monsieur le rapporteur. Vous avez dit qu'à partir du moment où ça n'est pas diffusé à la télévision ce n'est pas une action militante mais on ne vit pas au 19ème siècle maintenant désormais vous avez même des téléphones. Vous avez tout un tas de moyen de diffusion autre que la télévision. Donc ça, ça n'est pas tenable est ce qu'on est en train de faire ce soir. À minuit, un peu plus de minuit, on crée quand même des précédents assez dangereux. À travers ce type vous savez pas quel régime il pourrait y avoir plus tard dans notre pays mais dans les pays dans lesquels on interdit. Des activités militantes pacifique, ce ne sont pas des pays démocratiques et dans certains pays, il y a eu des Jeux olympiques, comme en Chine là bas effectivement, on n'a pas le droit de faire ça si c'est ça les modèles que vous prenez en prenant des mesures d'exception de ce type là, qui plus tard pour être reprise dans le droit commun pour tout un tout un tas d'autres événements, c'est très dangereux. Je pense que vous vous rendez pas compte des précédents, que vous êtes en train de créer.

J'ai quand même répondre à monsieur Chantrel, je n'ai pas parlé d'action militante. J'ai parlé de manifestations. Ce qui est différent. Et la conséquence de ces manifestations, c'est d'interrompre le cours du jeu sans que le SMIC téléspectateurs soit au courant de ce qui se passe. Merci monsieur le rapporteur. Alors je mets aux voix. L'amendement 11 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté un amendement 12 même avis même vote. Il n'est pas adopté le 13 même avis même vote. Il n'est pas adopté et enfin le 14 même avis même vote. Il n'est pas adopté, je mets aux voix l'article 12 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Alors Monsieur savant souhaite qu'on arrête la séance où vous souhaite présenter son amendement.

Rappelle que le fait de troubler le déroulement d'une compétition de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de biens en pénétrant sur l'aire de compétition d'une ancienne sportif. Peut être puni donc d'Alain d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Ces personnes encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendent aux abords d'une enceinte où se déroule donc une manifestation sportive au travers donc de l'article L 332 tirer 11 du compte du sport par contre le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement de la retransmission possible d'une manifestation sportive. Elle est puni de 7500 euros le fait pour l'auteur de cette infraction de se rendent coupables de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours et lui aussi puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Mais le juge ne peut prononcer la peine complémentaire qui est prévu dans le code du sport d'interdiction de du stade, mon amendement propose que cette peine complémentaire soit également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies, notamment l'article L 222 tiré 13 du code pénal qui prévoit que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou en entrée aucune incapacité de travail. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Avis de la commission. fait référence à l'article L 222 13 du code pénal qui liste les violences qui sont, puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, parmi lesquels figurent les violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation et celles réalisées dans un moyen de transport collectif de voyageurs. son amendement propose d'étendre la liste. De ces délits aux violences commises dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive. Cet ajout à l'article L 222 13 du code pénal semble justifiée, compte tenu des autres circonstances qui sont évoqués, néanmoins. Afin de s'assurer que cet ajout ne portera pas préjudice à la cohérence de notre droit pénal. Je, je souhaite connaître l'avis du gouvernement, sur cette disposition. Merci monsieur le rapporteur, madame la ministre. Avis du gouvernement. On partage évidemment hein le, l'objectif du sénateur ça hein de de faire cesser absolument toutes les formes de violence dans nos stades. Mais ce qui nous ennuie c'est la création d'une circonstance aggravante aggravante qui aurait en plus pour effet de élargir puisqu'il s'agit de de violences légères de manière très importante, très large. L'application de peines pour le coup, très importante, 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende. Donc cette proposition nous semble quelque peu disproportionné et ne permet pas un autre sens d'atteindre ce point d'équilibre qu'on a essayé de constamment préserver entre la sauvegarde de l'ordre public lors des grands événements et la proportionnalité de la peine. Merci madame la ministre, monsieur le rapporteur. Vous suivez l'avis du gouvernement. Donc, avis défavorable. Monsieur pour explication de vote.

Présent et des problématiques qui sont très présents dans les stades avec des violences récurrentes, aussi bien dans les tribunes que dans les travées que. Aller à proximité des stades, donc il y a urgence à à renforcer cette. Ce dispositif. Quand vous parlez. De peines légères mais on parle quand même d'incapacité de travail. Sur des personnes qui sont, qui subissent ces violences. Donc moi je fais confiance aussi à la justice de trouver le bon équilibre dans les sanctions, mais au moins qu'on puisse rajouter la possibilité au moins de l'interdiction de stade.

dans la l'impossibilité de revenir dans un équipement sportif, donc. Si vous voulez qu'on qu'on réponde à cet objectif de ramener de la sérénité de la tranquillité et la sécurité dans les stades ou des familles viennent avec des enfants qui se retrouve des fois au milieu d'agressions qui peuvent subir moi je trouve que l'interdiction de stade doit aussi. C'est un élément supplémentaire pour la justice. C'est pas une obligation mais le juge, au moins le juge aura la possibilité de l'appliquer. Aujourd'hui il peut pas l'appliquer. Merci cher collègue. Monsieur le Président la font. Vous avez la parole. moi je voudrais juste essayer de trouver une voie de passage pouvoir. Donner suite à la proposition de du du sénateur ça va j'ai entendu les, les réponses de la ministre qui dispose peut-être il y a. Un peu disproportionné par rapport au fait néanmoins ce texte soit acheminer entre l'Assemblée nationale et la CMP. Je pense que ça serait bien qu'on le laisse. Qu'on vote l'amendement du sénateur ça va et ce qui donnera le temps de de retravailler et bien sûr avec, avec vous, madame la Ministre si ça convient au rapporteur évidemment. À titre personnel j'émettrai un avis de sagesse. Merci monsieur le rapporteur. Et donc. Je vais mettre aux voix l'amendement 89 qui reçoit une sagesse de la commission Défavorable du coup du gouvernement qui est. Pour. Qui est contre. Qui s'abstient il était. Adopté la parole. Est à monsieur Jean-Pierre de colle pour une mise au point, au sujet d'un vote. pour le scrutin 111 le groupe les indépendants. Dans sa totalité votre contrat. S'il a été donné de votre mise au point ne sera publié au Journal officiel et figurera l'analyse politique du scrutin concernés j'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies. Renouvelables les parvenu à l'adoption d'un texte commun. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Nous avons examiné 32 amendements au cours de la journée, il en reste 23 examiner sur ce texte. Prochaine séance mercredi 25 janvier à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.